les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie mercredi 20 février sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- L'ordre du jour appelle la discussion en première lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli. Cette proposition de loi a été adoptée à la fin du mois de novembre à l'Assemblée nationale, et je me réjouis que la Haute Assemblée se saisisse désormais de ce texte. J'en suis d'autant plus heureux que j'ai eu à suivre ce texte comme député ; c'est donc avec une sincère émotion que je suis présent aujourd'hui pour représenter le Gouvernement. Il est impossible de ne pas ressentir une certaine émotion lorsque l'on évoque les cancers pédiatriques. Nous avons tous en mémoire ces visages d'enfants et la douleur inaltérable de leur famille. Le sentiment d'injustice est inhérent à la maladie, qui frappe aveuglément et brutalement. L'autre sentiment qui émerge lorsque l'on parle de ce sujet est celui de l'urgence : l'urgence de traiter, d'en sortir ; mais aussi l'urgence de développer de nouveaux traitements l'urgence de pouvoir accéder à un médicament ou à un essai clinique ; l'urgence de trouver pour guérir. Cette urgence a été bien comprise par Mme la rapporteur et par l'ensemble des sénateurs de la commission des affaires sociales, qui ont pris la responsabilité d'adopter à l'identique le texte de l'Assemblée nationale et de permettre ainsi une adoption conforme. Je les conforme. Je les en remercie. Le texte pourra entrer en vigueur rapidement. C'est tout ce que l'on doit collectivement aux enfants et à leurs familles. Néanmoins, j'ai entendu vos remarques et vos critiques sur le texte adopté par l'Assemblée nationale. Je souhaiterais prendre le temps de répondre à quelques-unes des réserves que vous avez pu exprimer.

Des parlementaires siègent dans toutes les agences sanitaires. C'est une bonne chose qu'il en soit de même à l'INCa. En revanche, un contingent de quatre parlementaires, tel qu'il est envisagé, aurait été excessif à nos yeux, avec le risque de déséquilibrer la composition du conseil d'administration de l'INCa. Aussi, il a été proposé de le limiter à deux parlementaires. Vous avez également émis des réserves sur la nouvelle rédaction de l'article 2, réserves que je peux entendre. Les travaux de la rapporteur à l'Assemblée nationale avaient indiqué que l'interprétation des dispositions du code de la santé publique par les comités de protection des personnes se révélait parfois être un frein. Nous avons entendu son souci de traduire les préoccupations des familles qui craignent que des enfants ne puissent participer à des essais cliniques. Aussi, nous avons souhaité qu'il apparaisse clairement à l'article L. 1121-7 du code de la santé publique que des recherches pédiatriques peuvent être réalisées. Cette nouvelle rédaction affirme ainsi la possibilité de faire des recherches pédiatriques tout en garantissant un haut niveau éthique et de sécurité à ces recherches. Sur la question de l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP, nous essayons de trouver des solutions. Je suis convaincu que cette proposition de loi permettra de procéder à une avancée significative pour les enfants malades et leurs familles. Mais vous avez raison cela ne nous empêchera pas de nous interroger sur l'articulation entre les différentes prestations existantes. Je pense ici à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, et à la prestation de compensation du handicap, la PCH enfant- certes, ce n'est pas une vraie PCH enfant à ce stade qui ont vocation à aider les parents ayant besoin soit de réduire ou d'interrompre leur activité professionnelle, soit de faire appel à une tierce personne, soit d'engager des frais pour s'occuper de leur enfant malade, avec une gamme d'aides plus large que l'AJPP, qui est concentrée sur la seule compensation de l'interruption d'activité.

Vous le savez, Agnès Buzyn s'est personnellement battue lorsqu'elle dirigeait l'INCa pour ce droit à l'oubli, sans lequel les anciens malades continuent à porter le fardeau de la maladie alors qu'ils essayent de concrétiser un projet de vie. Des travaux sont déjà engagés et évoquent la possibilité de déplacer la borne d'âge. Ils doivent- et vont -se poursuivre. Notre détermination collective ne peut pas être mise en doute.

malades, quel que soit leur âge. Il nous semble impératif de respecter le processus propre à la convention AERAS, qui continue de faire ses preuves, pour le plus grand bénéfice des patients.

Les groupes d'études des deux assemblées sont mobilisés de longue date sur ce sujet. Notre collègue Catherine Deroche nous a efficacement sensibilisés à cet enjeu, si bien que nous sommes nombreux à avoir soutenu à la fin du mois de janvier la demande d'un collectif associatif de déclarer la lutte contre les cancers pédiatriques grande cause nationale. Le Parlement est donc pleinement engagé. Nous comptons désormais sur l'action du Gouvernement et des industriels. Le texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale a le mérite de proposer une stratégie globale dans notre politique de lutte contre les cancers de l'enfant, de la relance de la recherche en oncologie pédiatrique à l'accompagnement social des parents, en passant par la prise en charge de la douleur et le droit à l'oubli des jeunes traités pour un cancer dans leur adolescence. Notre commission a salué cette démarche, tout en regrettant les imperfections de la proposition de loi. Les ambitions du texte ont en effet été revues fortement à la baisse par le Gouvernement. Les avancées effectives sont essentiellement au nombre de deux. La première consiste en la prise en compte de la recherche sur les cancers de l'enfant dans la stratégie portée par l'INCa, dont l'horizon temporel et les appels à projets subséquents ont été allongés, afin de tenir compte du temps long que nécessite l'inclusion des patients mineurs dans les essais cliniques. La seconde réside dans l'assouplissement des conditions du bénéfice du congé de présence parentale et de l'allocation journalière afférente. Ce sont des progrès dont l'ensemble des parties prenantes se félicitent. En revanche, notre commission a déploré plusieurs occasions manquées. Elle reste d'ailleurs déterminée à faire avancer les choses sur ces sujets à l'occasion de l'examen d'autres textes. Tout d'abord, l'article 2 avait le mérite de poser la question essentielle de l'accès des mineurs, en particulier des adolescents, aux essais cliniques de phase précoce. On sait que les industriels sont encore peu enclins à étudier la pertinence de thérapies innovantes chez les adolescents, en mettant en avant le principe d'interdiction générale d'inclusion des mineurs dans des essais cliniques si ceux-ci peuvent être menés avec une efficacité comparable chez les adultes. Ils font également valoir la dérogation du règlement pédiatrique européen de 2006, qui les dispense de plan d'investigation pédiatrique lorsque l'indication n'existe que chez l'adulte. Or les nouvelles thérapies ont la particularité de cibler des voies d'activation de tumeurs qui se retrouvent chez l'adulte comme chez l'enfant. La rédaction proposée par le Gouvernement et retenue par l'Assemblée nationale ne change en réalité pas l'état du droit en vigueur. Remplacer « ne peuvent que si » par « peuvent seulement si » a un effet purement lexical. La tournure est positive, mais le droit ne change pas, même si on peut y voir une volonté d'affichage. Sur le droit à l'oubli, l'Assemblée nationale a respecté le processus conventionnel qui préside à la convention AERAS. Nous nous en félicitons. Toutefois, le délai prévu n'est contraignant que pour l'ouverture d'une négociation. En ne fixant pas de délai pour la conclusion de cette négociation, le texte n'astreint pas les partenaires à une obligation de résultat. Nous pouvons comprendre une certaine prudence sur le sujet épineux de l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé. Nous resterons néanmoins particulièrement vigilants quant au déroulement de cette négociation. Par ailleurs, l'article 1 est problématique. Nous gravons dans le marbre la présence au conseil d'administration de l'INCa de parlementaires. Notre commission est réservée sur l'opportunité de cette disposition, qui alimente un mélange des genres, en plaçant des parlementaires potentiellement en situation de juge et partie d'un côté, ils participeront à une instance décisionnelle avec d'importants pouvoirs d'agrément et d'attribution de financements, et seront donc organiquement liés à la gestion de l'INCa ; de l'autre, ils contrôleront l'activité de l'institut, le Parlement devant, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, se prononcer sur son niveau de financement. Il nous appartiendra à l'avenir de mettre un terme à ce type de confusion. Sur le thème de la prise en charge de la douleur, la loi n'est sans doute pas le vecteur le plus opérationnel ; à notre sens, un nouveau rapport l'est encore moins. La prise en charge de la douleur est d'ores et déjà une priorité du développement professionnel continu des professionnels de santé. Là encore, les leviers d'actions sont entre les mains du Gouvernement et des industriels. D'une part, il appartient aux industriels de renforcer leurs efforts dans le développement d'antidouleurs adaptés, dans leur posologie et leur forme galénique, à l'enfant. Aujourd'hui, entre le paracétamol et la morphine, les alternatives font cruellement défaut. D'autre part, le Gouvernement doit donner aux centres de cancérologie pédiatrique les moyens de développer en interne une véritable coordination de la prise en charge de la douleur, afin de prévenir ou d'alléger sa chronicité et d'assurer la continuité de la prise en charge avec la médecine de ville. Les soins de support, en particulier l'accompagnement psychologique, doivent trouver toute leur place dans le parcours de soins des jeunes patients. Nous appelons à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie du suivi de long terme des personnes traitées pour un cancer dans leur enfance ou adolescence. Il s'agit non seulement de mieux gérer les conséquences des traitements sur la qualité de vie des jeunes adultes, mais également de garantir un suivi psychologique sur la durée. Les séquelles potentielles à l'âge adulte peuvent en effet se révéler lourdes et méritent d'être mieux anticipées insuffisance cardiaque ou rénale, complications thyroïdiennes, mais aussi, bien souvent, troubles psychologiques. Vous l'aurez compris, le texte n'est pas parfait et aurait pu faire l'objet d'améliorations. Chaque petit pas est précieux dans l'amélioration de la prise en charge des enfants et adolescents traités pour un cancer et de la situation de leurs parents. Les avancées proposées par ce texte doivent se matérialiser le plus rapidement possible, dans l'intérêt de la recherche en oncologie pédiatrique, sujet qui, je le sais, tient particulièrement à coeur à Mme la ministre des solidarités La commission a donc adopté sans modification la proposition de loi, et invite le Sénat à l'adopter définitivement dans les meilleurs délais. La parole

monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain votera la proposition de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli, malgré des reculs sérieux par rapport au texte initialement déposé à l'Assemblée nationale ; nous voulons répondre aux attentes des associations de parents, qui souhaitent une adoption rapide. À ce propos, je souhaite formuler une observation. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à une alternative un peu compliquée : voter conforme ou faire prendre du retard. voter conforme ou faire prendre du retard. Ce n'est pas une bonne alternative dans le cadre du travail parlementaire. Je sais bien que, en ce moment, il est de bon ton de critiquer le bicamérisme, et particulièrement le Sénat, mais notre Haute Assemblée a vocation à apporter davantage à l'élaboration législative qu'un vote conforme aux propositions de loi de l'Assemblée nationale. C'est bien vrai ! Nous regrettons en effet que la proposition de loi ait été en grande partie vidée de sa substance par des modifications apportées à l'Assemblée nationale par la majorité présidentielle, très probablement à la demande du Gouvernement. Sûrement ! Il est donc indispensable de poursuivre le travail engagé pour améliorer l'accompagnement des familles, renforcer le droit à l'oubli et faire progresser les conditions de la recherche. En particulier, nous ne sommes pas totalement convaincus par l'article 2, qui nous semble être essentiellement un article d'affichage. Il n'améliore pas le droit en vigueur des essais cliniques sur les mineurs, alors même que l'ouverture des essais cliniques constitue un enjeu important pour permettre une véritable adaptation des traitements aux enfants et aux adolescents. Les enfants et les adolescents doivent être considérés non pas comme des adultes miniatures, mais comme des patients à part entière, nécessitant une prise en charge spécifique. C'est pour cela que les essais cliniques sont cruciaux, et l'article 2 ne répond pas à ces enjeux. Nous aurions souhaité que cette proposition de loi soit plus ambitieuse, en matière de recherche bien sûr, mais également vis-à-vis des jeunes malades, puis des jeunes guéris, qui peuvent enfin retrouver une vie normale, sereine, en prenant peu à peu de la distance par rapport à la maladie. Il aurait fallu faire preuve de davantage de volontarisme vis-à-vis du droit à l'oubli, afin qu'il soit étendu aux jeunes âgés de dix-huit Le Gouvernement en a décidé autrement. Je le regrette d'autant plus qu'il s'agissait d'une promesse de campagne du Président de la République, qui déclarait : « Nous renforcerons le droit à l'oubli pour les personnes ayant été malades. Au moment de souscrire un emprunt ou un contrat d'assurance, les malades de cancers et de l'hépatite C n'auront plus à le mentionner dès cinq ans après leur rémission, contre dix ans aujourd'hui. Nous l'étendrons aussi à de nouvelles maladies. » C'était au mois de mars 2017. Deux ans plus tard, nous devons nous contenter pour l'instant d'une situation de compromis, par par le biais d'une négociation au sein de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Certes, les négociations sont utiles ; nous les apprécions beaucoup. Mais, dans cette maison, nous préférons, lorsqu'il s'agit des droits de la personne, la loi à la négociation. Nous nous réjouissons en revanche de la prise en compte de la durée totale de l'allocation journalière de présence parentale dans le calcul de l'ancienneté. Il s'agit là d'une avancée importante pour les aidants familiaux.

oui ! C'est une question de justice, puisque c'est limiter autant que faire se peut une détérioration des revenus du travail et des pensions de retraite. Cependant, de nombreuses progressions sont attendues pour que le rôle d'accompagnant soit facilité. Par exemple, aujourd'hui encore, pour celles et ceux qui habitent loin des centres de soins, la problématique de l'hébergement peut entraîner des frais importants pour les familles. La question ne doit pas être considérée comme réglée. Aujourd'hui, un petit pas est fait. Il est nécessaire d'aller plus loin. Nous souhaitons que le Gouvernement se saisisse plus fermement du sujet, afin que de véritables progrès soient effectifs, que nous fassions à l'avenir non plus de petites avancées, mais de grands pas dans la prise en charge des cancers pédiatriques. Le prochain plan Cancer doit prendre en compte les grands besoins de la recherche en cancérologie pédiatrique et, plus largement, les besoins de la recherche sur les maladies pédiatriques rares, notamment parce qu'il n'a pas été possible de favoriser la recherche l'article 2. Je pense que ce plan Cancer ne devra pas décevoir.

les chiffres sont connus, mais il est parfois bon de les rappeler, voire de les marteler, notamment sur un sujet aussi sensible que celui du cancer de l'enfant : 500 enfants meurent encore chaque année du cancer. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de quinze Pourtant, les cancers pédiatriques souffrent d'un déficit d'investissement dans la recherche et d'un accompagnement largement perfectible. Certes, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'a pas vocation à changer la face du monde. Mais elle offre néanmoins des avancées que je salue sans retenue. D'abord, la définition d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer permettra notamment de fixer un seuil minimal d'investissements publics destinés à la recherche pédiatrique. Cette stratégie, mise en oeuvre et évaluée à mi-parcours par l'INCa, nous est aujourd'hui indispensable et justifierait presque à elle seule le vote de cette proposition de loi. On sait que les trois plans Cancer successifs ont permis des avancées majeures. Chez l'enfant, le taux de guérison est passé de 50 % à 80 % depuis 2003. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L'investissement public paie. Depuis le projet de loi de finances pour 2019, un budget propre de 5 millions d'euros a été attribué à la recherche oncopédiatrique. Les associations espéraient 20 millions d'euros. Cette ambition peut paraître insuffisante. Mais, face au cancer d'un enfant, rien ne peut sembler à la hauteur. Néanmoins, cette avancée, couplée à celle de l'article 1, permettra certainement d'améliorer la situation ; nous l'espérons. Elle pourrait notamment attirer de nouveaux chercheurs, qui craignaient jusqu'ici de passer plus de temps à chercher des financements que de nouveaux traitements. Parmi les autres avancées figure la volonté d'améliorer l'accompagnement des malades et de leurs familles. Le cancer d'un enfant est toujours vécu comme une injustice- c'est une injustice ! -, comme un séisme au sein d'une famille entière. Améliorer l'accompagnement de l'enfant malade par ses parents est pour moi la moindre des choses que l'on puisse faire. L'article 3 permet ainsi d'adapter le congé et les allocations de présence familiale à la pathologie, à son évolution et à sa durée, comme l'ont souligné avec d'autres mots les auteurs de cette proposition de loi. Le réexamen de cette durée permettra notamment à la famille de rester auprès de l'enfant tout au long de la maladie et de faire face à une éventuelle rechute, que l'on sait malheureusement possible. Les articles 5 et 5 s'intéressent à une autre problématique tout aussi primordiale : le droit à l'oubli. La rédaction issue de l'Assemblée nationale invite les partenaires à engager une négociation, afin d'étendre à l'ensemble des pathologies cancéreuses, quel que soit l'âge, le droit à l'oubli cinq ans après la fin du traitement, pour retrouver l'accès au crédit et à l'assurance. Nous dépassons ici les frontières de l'oncologie pédiatrique, et c'est une bonne chose. Il s'agit d'une véritable bouffée d'oxygène pour ceux qui, après avoir subi un cancer, restent pénalisés dans leur quotidien et se confrontent à un vrai parcours du combattant à chaque nouveau projet de vie. Espérons que l'invitation à la négociation se concrétise dans les faits. Autre sujet d'importance : l'assouplissement des règles permettant à un enfant de prendre part à un essai clinique est une mesure essentielle pour faire avancer la recherche, notamment dans le domaine des traitements, pour les rendre plus performants, mais, surtout, moins toxiques. La préservation d'un haut niveau de sécurité et d'éthique ne doit pas en ce domaine freiner la recherche. Faciliter les conditions d'accès des enfants aux essais cliniques est plus que souhaitable. Comme l'a expliqué Mme la rapporteur, deux freins subsistent pour faire progresser la recherche : d'une part, les restrictions permettant à un mineur de participer à un projet de recherche ; d'autre part, l'étroitesse des populations concernées- c'est heureux ! -pour chaque pathologie. En effet, ce sont environ 2 500 jeunes qui sont concernés chaque année. Ce faible volume explique la frilosité des industriels, qui peinent à investir dans la recherche de traitements adaptés. Or la soixantaine de cancers pédiatriques qui se rapprochent davantage des maladies rares que des cancers de l'adulte, exige des stratégies thérapeutiques ciblées. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des conditions de traitement actuelles, dont l'adaptation de traitements destinés aux adultes peut entraîner- je l'ai déjà souligné -de lourdes conséquences sur la santé à long terme. La rédaction retenue par les députés pour cet article 2 ne change en rien l'état du droit en vigueur ; on peut le regretter. Elle démontre une ambition, une voie à suivre. Nous espérons qu'elle portera ses fruits dans un avenir proche. L'investissement financier de l'État, à hauteur de 5 millions d'euros, est un premier acte concret. Il faudra certainement s'interroger de nouveau sur les règles qui régissent aujourd'hui l'accès des mineurs aux essais cliniques. Le Gouvernement a proposé un amendement, devenu article 2 , qui vise à étendre de cinq ans à huit ans la durée des appels à projets de l'INCa, afin de tenir compte du temps plus long de l'inclusion dans la recherche clinique chez l'enfant. Sur ce point, je fais confiance à la ministre, ou plutôt à la spécialiste, et je soutiens cette proposition. Des doutes subsistent néanmoins sur les articles 1 et 4 . Comme d'autres, je ne suis pas certaine que la place des parlementaires soit au conseil d'administration de l'INCa. Nous avons bien d'autres moyens de contrôle de ses objectifs. de contrôle de ses objectifs. Le groupe du RDSE n'est généralement pas favorable aux demandes de rapport. Toutefois, la prise en charge de la douleur doit faire partie des priorités de ce gouvernement. Cela fait maintenant trop longtemps que le sujet revient sur la table sans que sa prise en charge soit encore optimale, ni chez l'enfant ni chez l'adulte. Et de grandes disparités territoriales persistent. En effet, la question de la formation des professionnels sur la prise en charge de la douleur ne relève pas du domaine de la loi. Je formule donc le souhait qu'un tel rapport, s'ajoutant aux nombreux autres constats de carence dans le domaine de la douleur et des soins palliatifs, débouche enfin sur des mesures efficaces. efficaces. Le groupe du RDSE, malgré ces quelques réserves, soutient l'esprit général du texte. Désireux d'en voir les dispositions rapidement mises en oeuvre, ses membres voteront en faveur de son adoption conforme.

Qu'il s'agisse de la leucémie, cancer le plus fréquent chez l'enfant, du cancer du système nerveux central, des lymphomes ou d'autres formes, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants. Pourtant, la médecine a fait des progrès importants dans le traitement des cancers. À l'époque où la majorité d'entre nous étaient encore enfants, seulement une personne malade sur cinq en guérissait. Actuellement, après trois plans Cancer successifs, quatre enfants sur cinq en guérissent, mais, malheureusement, 500 enfants meurent encore chaque année à la suite d'un cancer. Les cancers pédiatriques, très différents des cancers de l'adulte, ne disposent que rarement de traitements spécifiques. Le plus souvent, ils sont traités en adaptant des doses de chimiothérapie pour l'adulte, selon le poids et l'âge du jeune patient. Aussi, le développement de la recherche en oncologie pédiatrique, principale mesure proposée par ce texte, est primordial pour favoriser la guérison, mettre en place de nouvelles thérapies et limiter le risque de rechutes et de séquelles laissé par les traitements. Le déploiement d'une stratégie nationale de coordination de la recherche est une première étape importante

mais devrait permettre aux enfants, lorsque c'est pertinent, de recevoir des traitements innovants afin d'éviter toute perte de chance. L'article 2 tend à allonger la durée limite des appels à projet lancés par l'INCa à huit ans au lieu de cinq ans, ce qui est pertinent. Une autre disposition très importante de cette proposition de loi est l'adaptation du plafonnement de l'allocation journalière de présence parentale à la durée réelle de la maladie. Cela contribuera à améliorer le quotidien des familles et l'accompagnement de leur enfant. L'article 4

dès cinq ans après la rémission au lieu de dix ans. Cette mesure représente une avancée supplémentaire vers l'égalité, limite la double peine et offre la possibilité aux anciens malades d'envisager l'avenir après leur maladie. Mais, à cet âge, attendre cinq ans après la guérison

Au-delà de l'amélioration des traitements, qui est capitale, quelle politique de prévention mettre en place pour limiter les facteurs de risques ? Ces chiffres laissent une grande incertitude quant à l'origine de 90 % des cancers. Les chercheurs ont établi que la fenêtre d'exposition au risque est plus importante au cours de la vie foetale et dans la petite enfance. Cela est dû à une vulnérabilité dans la mutation des gènes, à un métabolisme hépatique limité, ou à une absorption élevée du toxique associée à une forte prolifération cellulaire au cours de ces périodes critiques du développement. En conséquence, le déploiement d'une politique de prévention nous paraît utile afin de lutter efficacement contre les cancers, en identifiant, si possible, les facteurs de risque pour mieux prévenir l'exposition des des populations les plus vulnérables et ainsi limiter le déclenchement des cancers. Notre groupe a proposé en commission un amendement d'appel visant à inscrire la prise en compte des facteurs de risque liés au mode de vie et à l'environnement au sein des missions attribuées à l'INCa. secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour objectif de réunir les conditions d'une politique ambitieuse de prise en charge globale, sociale et médicale, d'oncologie pédiatrique dans les huit ans à venir. Nous savons que celle-ci doit être votée conforme pour une application rapide. Vous avez notre soutien. La

Milon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, légiférer sur les cancers pédiatriques nous rappelle que rien, dans la vie, ne prépare les familles à affronter l'annonce d'un cancer ou d'une maladie grave, d'autant plus lorsqu'elle touche un enfant. Chaque année, en France, 2 500 enfants ou adolescents doivent repousser leurs limites face à la maladie. Chaque année, près de 500 familles sont endeuillées par le décès d'un enfant ou d'un adolescent des suites d'un cancer. Malgré les progrès de la recherche, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d'un an. Mon collègue Jean-François Rapin développera plus particulièrement le volet concernant l'accompagnement des familles. Je centrerai mon propos sur la recherche en oncologie pédiatrique qui a été l'objet du colloque intitulé « Pour accélérer le développement de traitements spécifiques pour les enfants atteints de cancer », qui s'est tenu samedi dernier au Sénat sous le parrainage de notre collègue Catherine Deroche- j'en profite pour saluer son engagement plein et entier pour cette noble cause. Ce colloque organisé depuis plusieurs années par l'association a mis notamment l'accent sur l'importance de l'accès précoce aux médicaments innovants et sur les enjeux et les perspectives de la recherche. Les cancers de l'enfant ne sont pas similaires à ceux de l'adulte. Ils méritent donc un traitement spécifique. Ils sont plus rares et moins nombreux. Un tiers des cancers pédiatriques n'existent pas chez les adultes et, inversement, plus de 80 % des cancers de l'adulte ne se retrouvent pas en pédiatrie. Le développement

les laboratoires pharmaceutiques à développer une forme pédiatrique pour tous les nouveaux médicaments. Les effets de cette réglementation commencent à se faire sentir, les domaines dans lesquels le plus grand nombre de plans d'investigation pédiatrique achevés ont été enregistrés sont l'immunologie et la rhumatologie, pour 14 %, les maladies infectieuses, pour 14 %, les maladies cardiovasculaires, pour 10 %, et les vaccins, pour 10 % L'oncologie a les moins bons résultats en ce qui concerne le nombre de plans d'investigation pédiatrique approuvés, ne représentant que 7 % des plans d'investigation achevés. En France, la création de centres labellisés INCa de phase précoce a été lancée en 2010. Des infrastructures sont financées afin d'accélérer les innovations pour les enfants en échec thérapeutique. Grâce à cette démarche, les efforts de structuration de la recherche clinique de phase précoce se poursuivent. Actuellement, sur les seize centres labellisés, six ont une activité de phase précoce en cancérologie pédiatrique. À l'échelle internationale, la France participe à 13 % des essais pédiatriques et à 19 % des essais oncopédiatriques. Afin de sensibiliser, mobiliser et développer les initiatives « pour guérir plus et guérir mieux les cancers de l'enfant », l'Institut Gustave-Roussy a lancé en France le mouvement Septembre en or. La recherche de notre pays en cancérologie pédiatrique est donc active et de très grande qualité. À cet instant, je tiens à rendre hommage au travail et à la détermination des équipes de chercheurs et de soignants qui persévèrent chaque jour pour développer de nouvelles armes thérapeutiques. Pourtant, des freins au développement de la recherche existent Notre collègue Jocelyne Guidez, dont je tiens à saluer la qualité du travail, pointe l'un des freins au développement des essais cliniques. Les professionnels de santé, les chercheurs et les associations de patients et de parents déplorent les contraintes d'âge pour l'inclusion de mineurs dans des essais cliniques. Le centre SIREDO de l'Institut Curie a également souligné que, si les projets multicentriques internationaux sont élaborés par des comités d'investigateurs experts et évalués par des experts extérieurs, persiste le problème de l'accès aux nouveaux médicaments hors essai, parfois non accessibles aux adolescents, y compris en autorisation temporaire d'utilisation, ATU. L'article 2 de la proposition de loi est probablement une amélioration d'un point de vue juridique, mais il ne va pas assez loin dans l'inclusion de patients mineurs dans des essais cliniques. J'ose dire que cet article relève plus d'une « volonté d'affichage » que d'une volonté d'efficacité. Par ailleurs, l'un des enjeux des plans Cancer successifs est d'élargir l'activité de recherche au plus grand nombre possible de centres. Les parents des jeunes patients ne sont pas tous mobiles, ils n'ont pas forcément la possibilité ou les ressources pour répondre à toutes les contraintes d'un essai lorsque celui-ci se déroule dans un centre situé loin de leur domicile. Si nous souhaitons que davantage de patients participent aux essais, il est indispensable d'apporter la recherche à proximité des patients. J'en viens à la participation des parlementaires au conseil d'administration de l'INCa. Nous trouvons cette mesure inappropriée. Nous soutenons l'avis de la rapporteur quant à la création d'un mélange des genres plaçant les parlementaires en situation de « juge et partie » ; ces derniers sont en effet chargés de contrôler la gestion de l'INCa et de voter son budget à l'occasion du projet de loi de finances, et non pas de juger du bien-fondé de certaines recherches. Enfin, les trois articles ayant pour objet des demandes de rapports ne nous satisfont pas ; c'est une tradition au Sénat. Ils sont superfétatoires : les données demandées existent déjà soit dans des rapports d'activité, soit dans des rapports d'évaluation. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains estime que ce texte aurait pu être amendé et certainement amélioré avec les précisions que notre collègue Jocelyne Guidez souhaitait apporter. comme nous avons compris que les modifications qui pourraient être introduites par le Sénat mettraient en péril le devenir de cette proposition de loi, dans l'intérêt des jeunes malades, nous la voterons conforme.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, en 2017, pendant plusieurs mois, un immense portrait a été placardé sur la tour Montparnasse : celui de Noé décédé d'un cancer à l'âge de dix ans. En dessous de ce portrait, il y

En outre, la fréquence des cancers chez les enfants de moins de quatorze ans a augmenté de 13 % entre les années 1980 et 2000. Des chiffres qu'on voudrait ne plus entendre. Ceux qui, grâce à la science, guérissent gardent généralement des séquelles liées à la radiothérapie et à la chimiothérapie, et pour cause. Les cancers pédiatriques ont leurs spécificités propres et leurs origines sont encore mal connues. Coordonner la recherche sur les cancers pédiatriques, améliorer la situation des familles et la formation du personnel soignant sont les grands axes qui animent cette proposition de loi. Bien évidemment, l'Assemblée nationale a adopté ce texte à l'unanimité, et je sais que les neuf articles qui la composent font consensus dans notre chambre. De ce fait, permettez-moi d'en reprendre les faits saillants. L'article 1 impose à l'INCa l'élaboration d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer. L'article 2 permet une recherche clinique sur les mineurs- elle n'était jusqu'alors possible que sur les adultes -, tout en garantissant un haut niveau éthique et de sécurité à ces recherches. À l'article 2 , alors que les appels à projet de recherche ne pouvaient porter que sur des projets de cinq ans, ils peuvent désormais être faits sur des projets de huit ans. L'article 3 étend l'aide à l'accompagnement des parents sur toute la durée du cancer du mineur, alors À l'article 4 , il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport sur le traitement de la douleur des mineurs dans le cadre des soins qu'ils reçoivent. L'article 5 portait initialement sur le droit à l'oubli, à savoir la non-déclaration d'un cancer survenu antérieurement à la demande d'emprunt, sous certaines conditions. Les débats ont été très nourris à l'Assemblée nationale sur cette question. Je remercie Mme Buzyn d'avoir redit son engagement à ce sujet à cette occasion. Je la cite : « Je me suis personnellement battue pour ce droit sans lequel les malades continuent à porter le fardeau de leur maladie. » Il n'est plus possible d'alimenter par l'attente l'impatience et l'inquiétude des parents. C'est pourquoi nous avons pris bonne note que, si les négociations n'aboutissaient pas dans un délai de six mois, le Gouvernement fixerait par voie réglementaire ce « droit à l'oubli Monsieur le secrétaire d'État, nous savons votre attachement à cette question et c'est pourquoi nous comptons sur vous. À l'article 5 , il est demandé un rapport au Gouvernement sur l'accès à l'emprunt d'une personne ayant eu un problème grave de santé, cancer pédiatrique inclus. À l'article 5 , il est demandé un rapport au Gouvernement sur le financement de la recherche sur les cancers des mineurs. Nul ne doute que des modifications auraient pu parfaire ce texte,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant de discuter du contenu de la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe Union je souhaite revenir un instant sur le sort du seul amendement que nous avions déposé et qui a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. J'attire votre attention, mes chers collègues, sur cette irrecevabilité et sur un raisonnement qui remet en question notre droit fondamental d'amender les textes de loi. Notre amendement visait à créer une contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques afin d'augmenter les moyens de l'INCa, notamment pour la recherche sur les cancers pédiatriques, ce qui, vous en conviendrez, ne serait pas un luxe La commission des finances l'a déclaré irrecevable pour la raison suivante : parce qu'il « crée une contribution prélevée sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques dont le produit serait affecté à l'INCa, opérateur de l'État dont le financement est quasi exclusivement issu de subventions pour charge de service public, cet amendement a pour objet d'augmenter la capacité à dépenser de l'INCa et crée donc une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. » Autrement dit, notre amendement a été « retoqué » au motif que l'augmentation des moyens de l'INCa conduirait inévitablement à l'augmentation des dépenses de l'institut. Ce raisonnement n'a ni queue ni tête ! Ainsi donc, les moyens créeraient les besoins ? Remarquez, c'est le raisonnement qu'ont défendu les gouvernements successifs depuis des dizaines d'années, notamment en matière de santé, et que vous poursuivez, monsieur le secrétaire d'État, en limitant l'offre de soins.

J'alerte solennellement l'ensemble des groupes politiques présents dans l'hémicycle sur la restriction en cours du droit des parlementaires, ... Elle a raison ! ... d'autant que cette décision va dans le sens de l'intimation qui nous a été signifiée de voter ce texte conforme. Attention, mes chers collègues, cette remise en cause du droit d'amendement renforce celles et ceux qui pensent qu'il faut supprimer le Sénat, et qui sont convaincus de l'inutilité des parlementaires que nous sommes. Évitons de tendre le bâton pour nous faire battre

Actuellement, le cancer est un fléau qui touche 2 500 enfants et adolescents par an, dont 500 décèdent. Si les cancers demeurent des maladies rares chez ces jeunes, tandis que, chez les adultes, 400 000 nouveaux cas sont déclarés par an, il existe une soixantaine de cancers pédiatriques différents, dont les origines, le développement et les manifestations ont peu à voir avec ce que l'on connaît des cancers qui touchent les adultes. Cette spécificité justifie la sanctuarisation d'un budget pour la recherche sur les cancers pédiatriques. En France, jusqu'à cette année, seulement 3 % du budget de l'INCa étaient dépensés pour les enfants. les associations estiment le besoin de financement de la recherche en oncologie pédiatrique entre 18 et 20 millions d'euros. Le Gouvernement a été contraint de faire un geste en ajoutant 5 millions d'euros au budget de l'INCa dans la loi de finances pour 2019, mais nous ne sommes pas encore au niveau demandé par les associations.

Le texte coordonne autour de l'INCa la recherche en cancérologie pour fixer un plan quinquennal en faveur des cancers pédiatriques. Pour faire avancer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, l'article 2 prévoit de faciliter la participation des mineurs aux essais cliniques. Dans le même temps, nous sommes sensibles aux garanties fixées par la proposition de loi, tant la chronique a été défrayée par des accidents parfois dramatiques survenus chez des adultes. Ainsi, il est prévu que la participation des mineurs à des essais cliniques se fera sous la vigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des comités de protection de personnes. Permettez-moi d'être dubitative quant aux possibilités de cette agence à qui l'on demande toujours plus avec toujours moins

revanche, nous soutenons la proposition de déplafonner la prestation afin de couvrir la pathologie dans son intégralité, ce qui va dans le sens de la bataille de l'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer ou de leucémie en faveur de la revalorisation de l'allocation journalière de présence parentale. La proposition de loi prévoit également d'assouplir les conditions de bénéfice du congé de présence parentale et de l'allocation journalière afférente, en tenant compte de la durée et des conséquences des traitements, ce qui est un progrès par rapport à la situation actuelle. Nous regrettons néanmoins la suppression par la majorité gouvernementale, à l'Assemblée nationale, des articles prévoyant d'intégrer les cancers pédiatriques dans le processus de formation continue des professionnels et d'étendre le droit à l'oubli aux jeunes âgés de dix-huit ans à vingt et un ans, cinq ans après leur rémission contre dix ans aujourd'hui. Nous regrettons enfin que le texte ne prévoie pas de dispositions relatives au financement d'études sur les facteurs environnementaux dans la survenue d'un cancer chez l'enfant. Malgré ces limites- et je veux remercier notre rapporteur Jocelyne Guidez ainsi que Catherine Deroche pour la qualité de leur travail notre groupe votera cette proposition de loi qui permet une amélioration de la recherche en cancérologie pédiatrique et apporte un soutien aux patients et à leurs familles. La parole

lancée par ses parents, M. et Mme Blanc, à la suite du décès de leur fille atteinte d'une tumeur au cerveau ; sept ans après sa création, cette association a collecté 7 millions d'euros pour aider la recherche. Samedi dernier, au lendemain de la journée internationale du cancer de l'enfant, le Sénat accueillait le colloque FAST sur la recherche, rendez-vous annuel depuis six ans.

À tout juste seize ans, après le décès de sa grand-mère frappée d'une leucémie, elle avait créé l'association Aïda pour inviter les jeunes à s'engager en faveur des enfants malades. Ces associations naissent, le plus souvent, en réaction à la perte d'un être cher, et ces témoignages nous marquent indéniablement. En cet instant, je veux remercier notre collègue Catherine Deroche, qui s'investit depuis longtemps dans la lutte et qui a donné l'impulsion, en 2016, à la création d'un groupe d'études au Sénat. Elle nous invitait, il y a quelques semaines, à suivre le collectif d'associations Gravir pour déclarer la lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent grande cause nationale pour 2019. Ces actions citoyennes, fortes et justes, trouvent un légitime écho dans la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Je m'en réjouis et remercie notre collègue députée Nathalie Elimas de son travail. Notre rapporteur Jocelyne Guidez a lancé une série d'auditions auprès des représentants institutionnels, des professionnels de la santé et de la recherche, des associations, du secteur des banques et assurances. La proposition de loi aborde largement la problématique du cancer pédiatrique. La preuve en est le titre donné au texte, qui peut paraître un peu long, mais dont l'intention est toutefois très claire. Pêle-mêle, voici ce que j'ai pu relever de ces entretiens. Contrairement à ce que pense l'opinion publique, on avance ! » On retrouve le même état d'esprit sur le site d', qui annonce des avancées significatives depuis le dernier colloque, et cite la procédure accélérée de l'ANSM dédiée aux médicaments innovants, la la revue du tirage au sort des comités de protection des personnes, le fonds de 5 millions d'euros supplémentaires accordé par le ministère de la recherche et, enfin, des traitements de plus en plus personnalisés. Les cancers des moins de quinze ans représentent 0,5 % des nouveaux cas de cancers. Au vu de sa prévalence, le cancer pédiatrique peut être assimilé aux maladies rares qui nécessitent des traitements spécifiques. Un travail à l'échelle européenne est nécessaire afin de mieux identifier les types de cancer. Mais aujourd'hui c'est compliqué, chaque pays ayant ses propres normes ». « C'est pourtant un enjeu, à l'heure du et de l'intelligence artificielle. « Ces trente dernières années, d'énormes progrès grâce à la recherche clinique sont à noter. Maintenant, il faut aussi aller sur la recherche fondamentale. » Cela permettra la compréhension et la connaissance des phénomènes naturels, l'élaboration de théories ou de modèles explicatifs. explicatifs. « Les services de pédiatrie travaillent contre la douleur, mais le manque de moyens est notable. Les oncopédiatres se forment sur le terrain, d'une part, en raison du coût des formations et, d'autre part, parce que l'approche multipartenariale est intéressante. Les professionnels ont de grandes compétences techniques, mais ils souhaiteraient une formation initiale et continue plus structurée et plus adaptée, sur la prise en charge de la douleur notamment. Et puis encore : « Des psychologues arrivent dans nos services, mais leur nombre est insuffisant. Et lorsque l'on veut poursuivre le suivi auprès de l'enfant après son hospitalisation et auprès de sa famille, la prise en charge n'est pas remboursée. Le suivi psychologique pendant et après une maladie est pourtant utile dans l'accompagnement global et pour une totale résilience. Je pourrai encore citer beaucoup de propos échangés avec nos interlocuteurs. Le sujet des cancers pédiatriques est une question qui dépasse tous les corporatismes professionnels.

L'article 1 prévoit la présence au sein du conseil d'administration de l'INCa d'un député et d'un sénateur. Le Parlement contrôlant, la loi de finances, la gestion de l'Institut, les parlementaires siégeant se retrouveront juge et partie, comme l'a dit le président de la commission

L'article 4, enfin, est supprimé. L'auteur du texte proposait de renvoyer à un décret le soin de fixer le contenu des actions de formation du développement personnel continu, notamment pour ce qui concerne la prise en charge de la douleur ou le suivi psychologique, jugés insuffisants aujourd'hui. La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, s'est engagée « à ce que la formation à la douleur, notamment à la douleur pédiatrique, fasse partie des priorités de l'année 2019

L'ossature centrale de la proposition de loi, elle, demeure. Il s'agit des articles 1, 3 et 5. L'article 1 prévoit une élaboration collégiale de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, dans laquelle une part des crédits publics sera affectée à la recherche en cancérologie pédiatrique. Les enjeux de santé nécessitent de dresser un horizon lisible pour tous. Cet article pérennise la lutte contre le cancer. Ensuite, la proposition de loi a le mérite de ne pas rester circonscrite aux seules questions médicales. Elle a pour ambition d'embrasser plus globalement son sujet grâce à ses articles 3 et 5. Le texte s'inscrit dans le processus de mutation du parcours de soins vers le parcours de santé du patient.

Enfin, dans cette nouvelle logique de parcours de santé, il faut intégrer la question de l'après-maladie. Le droit à l'oubli fait partie des grandes avancées sociales de notre pays. C'est une question de justice. Mme Elimas avait pour ambition d'étendre ce droit à l'oubli aux jeunes âgés de dix-huit à vingt et un ans, dès cinq ans après leur rémission, contre dix ans aujourd'hui. C'était l'objet de l'article 5. L'Assemblée nationale a su maintenir son esprit, tout en respectant le processus de la convention AERAS. En conclusion, même si je regrette la moindre portée de ce texte, je salue l'initiative, l'esprit de nos débats et l'intérêt porté à ce sujet, aux enfants atteints de cancer et à leurs familles.

Si, comme moi, vous avez été confronté professionnellement à cette situation dramatique, angoissante et parfois désarçonnante, vous comprendrez mon désespoir de ne pas pouvoir agir assez vite, mieux, et avec des moyens et des avancées proportionnels à la détresse engendrée pour les parents, les frères et soeurs, la famille et les proches. Malgré de grands progrès, ces cancers restent la première cause de maladie chez l'enfant. Il est donc essentiel de mieux traiter cette maladie qui touche 1 700 d'entre eux chaque année. À cet égard, je salue l'initiative de mon collègue député Bernard Perrut qui a souhaité voir reconnaître le cancer pédiatrique grande cause nationale 2019. Le 4 février dernier, lors des rencontres de l'INCa, Mme la ministre de la santé a déclaré que 5 millions d'euros supplémentaires seraient alloués à l'oncopédiatrie.

une opération visant à ce que chaque parlementaire s'engage en faisant un don personnel de 1 000 euros afin d'intégrer un plus grand échantillon d'enfants aux recherches. Le résultat fut mitigé, mais l'essentiel est que l'on ait mis réellement le sujet sur la table et sensibilisé pleinement nos collègues.

ou de handicaps nécessitant des soins lourds et un accompagnement renforcé. Par ailleurs, l'article 5 prévoyait que le droit à l'oubli soit étendu aux jeunes âgés de dix-huit ans à vingt et un ans, dès cinq ans après leur rémission, contre dix ans aujourd'hui. Il s'agissait, me semble-t-il, d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Néanmoins, le Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction de l'article imposant une renégociation de la convention nationale AERAS, afin qu'elle mette en place ce fameux droit à l'oubli de cinq ans pour les jeunes atteints de cancer au-delà de Le groupe Les Républicains est favorable à cette avancée. Néanmoins, comme l'a souligné mon collègue Alain Milon, je regrette que le Sénat ait été contraint de voter conforme ce texte. En effet, je suis intimement convaincu du rôle de notre chambre dans le débat démocratique, trop souvent remis en cause ces derniers mois. D'autres avancées sont à envisager afin de gérer au mieux les enfants malades ainsi que leurs familles. Je pense notamment à la nécessité d'améliorer la pédagogie et l'accompagnement lorsque le diagnostic est posé. Les associations de patients ont une place prépondérante dans cette situation- Élisabeth Doineau vient de l'évoquer -et il est essentiel de pouvoir les soutenir dans ces démarches. Puisqu'il a été difficile d'amender ce texte, j'espère que le débat sera poursuivi lors de l'examen prochain du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation de notre système de santé. Dans cette attente, comme l'a annoncé le président Milon, mon groupe votera cette proposition de loi. La parole

elle se prénommait Éva. C'était une petite fille de sept ans et demi, pleine de vie, en parfaite santé, intelligente, pétillante et sportive. Rien ne laissait présager son destin tragique. Éva fait partie de ces 500 enfants et adolescents emportés chaque année par la terrible maladie du cancer. Mais que représentent ces 500 décès d'enfants face aux 150 000 que l'on dénombre annuellement chez l'adulte ? Une sorte de maladie rare. Rare parce que la prévalence est d'un cas pour 400 enfants ; rare également parce que les cancers pédiatriques, une soixantaine environ, sont très différents de ceux de l'adulte, surviennent très tôt et se développent sur une période relativement courte. Le résultat, nous le connaissons : des thérapies peu adaptées, dérivées de celles des adultes, je pense en particulier aux chimiothérapies, avec tous les risques que de tels soins comportent pour les enfants. Les études le démontrent : les adultes précédemment traités pour un cancer pédiatrique ont une qualité de vie affectée par les effets secondaires des thérapies et ils risquent un décès prématuré. Alors oui, il est urgent pour le législateur d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement des cancers de l'enfant et de faire souffler un vent d'espoir chez les malades et leurs familles durement éprouvées. Voici encore l'histoire de Guillaume : pendant plusieurs semaines, malgré trois visites aux urgences pédiatriques en Essonne et à Paris, aucun diagnostic n'est posé face à ses douleurs au genou, sa petite fièvre et sa perte d'appétit. Une rhumato-pédiatre d'un grand hôpital parisien, après un appel du généraliste qui s'alarme, les reçoit dès le lendemain. Elle va trouver le diagnostic en vingt-quatre heures : cancer osseux parti du fémur. La chimiothérapie adjuvante marchera bien au début. Mais le cancer de Guillaume va récidiver pendant la dernière des neuf chimiothérapies prévues. Et là, tous le savent- médecins, parents -, il n'y a pas de « solution Aujourd'hui, Guillaume a laissé à la recherche, grâce au programme Mappyacts, le profil moléculaire de sa tumeur particulièrement agressive et ses cellules souches. Ses parents rêvent qu'il ait laissé les clés pour sauver des enfants. Mais, pour cela, il faut soutenir la recherche fondamentale. La loi de finances pour 2019 a montré la voie en inscrivant un financement de 5 millions d'euros, pour coordonner l'engagement de plusieurs dizaines de chercheurs en pédo-oncologie. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est de nature à répondre aux enjeux de cette mobilisation, qui doit s'amplifier dans le sillage des plans Cancer successifs. En faisant de l'Institut national du cancer le pivot d'une stratégie globale de lutte contre les cancers pédiatriques, coordonnée avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés, les professionnels de santé et les patients, ce texte va dans le bon sens et permet d'envisager enfin les financements adéquats au développement de nouvelles thérapies spécifiques. Je me réjouis aussi de la mesure de déplafonnement adoptée concernant la durée maximale d'allocation journalière de présence parentale. Elle permettra de répondre aux attentes des familles accompagnant un enfant dont la grave pathologie nécessite une présence soutenue et des soins souvent très contraignants. Permettez-moi enfin de rappeler combien il est nécessaire que les anciens malades bénéficient d'un droit à l'oubli effectif. La maladie est une épreuve suffisamment lourde pour ne pas ajouter au combat des patients pour leur survie, une nouvelle épreuve consistant à quémander le droit d'emprunter, ou de s'assurer correctement, des années après leur guérison. Je l'ai vécu à titre personnel à trente ans : après un cancer très lourd, il n'était pas normal que des banques ou assurances puissent répondre, au moment où l'on souhaite mordre la vie à pleine dent et réaliser un projet immobilier : « Chère madame, vous resterez une personne à risque toute votre vie Certes, une loi a enfin été promulguée pour réparer cette injustice, mais il n'est pas rare encore- je le vois dans mon entourage -d'avoir des difficultés pour emprunter après cette maladie. C'est pourquoi j'approuve sans réserve les dispositions de la proposition de loi qui engage les signataires de la convention nationale AERAS à ouvrir rapidement une négociation, pour que s'applique à l'ensemble des pathologies cancéreuses le délai de cinq ans au-delà duquel aucune information médicale, relative à ces maladies survenues avant l'âge de dix-huit ans, ne peut être recueillie par les organismes assureurs. Certes, ce texte était perfectible et il aurait été judicieux de laisser au Sénat la possibilité de l'amender. Toutefois, dans l'intérêt des patients et pour engager sans tarder l'ensemble des acteurs à se mobiliser, nous le voterons dans sa version issue de l'Assemblée nationale. Enfin, je soutiens, monsieur le secrétaire d'État, la demande de très nombreuses associations de voir les cancers pédiatriques devenir grande cause nationale en 2020. La parole

j'ai bien entendu leurs différentes interventions. Je veux vous dire que cette proposition de loi s'intègre dans une stratégie globale et qu'elle ne répond évidemment pas à tous les problèmes. Comme certains d'entre vous l'ont souligné, les plans Cancer successifs ont permis des avancées dans le traitement et l'accompagnement des patients et de leurs familles. En matière de recherche, les centres d'essais cliniques de phase précoce, le programme AcSé- accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes -, le programme intégré de pédiatrie de l'INCa et, plus globalement, cet environnement favorable à l'innovation en France, comme vous l'avez souligné, monsieur le président Milon, avec les ATU ou encore le, vont être renforcés par les 5 millions d'euros supplémentaires que nous avons accordés dans la loi de finances. Mais nous sommes déterminés à aller plus loin plus loin encore. La ministre l'a annoncé récemment aux Rencontres de l'INCa, il faudra renforcer notre effort pour lutter contre les cancers de mauvais pronostic, en particulier pour les enfants et les jeunes, grâce à la recherche fondamentale pluridisciplinaire et au renouvellement de la recherche clinique avec des essais adaptés à de petits nombres de patients. Pour conclure, la lutte contre les cancers pédiatriques est une priorité pour l'ensemble du Gouvernement- je pense que vous n'en avez pas douté. Je m'exprime ici au nom d'Agnès

La séance est reprise.

L'ordre du jour appelle la discussion en première lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

ce n'est un secret pour personne : les appels téléphoniques intempestifs et répétés constituent une nuisance pour nos concitoyens. Nous en avons tous déjà fait au moins une fois l'expérience.

Au moment où s'ouvre la discussion en séance, je voudrais simplement insister sur le besoin de trouver une solution équilibrée entre le bien-être des consommateurs et la préservation des emplois dans les centres d'appels téléphoniques. Le démarchage téléphonique est un sujet complexe, non seulement pour ses aspects techniques, mais aussi par les risques d'impact sur l'emploi. Nous devons aborder la question avec beaucoup de soin. Tout l'enjeu est là : mieux protéger les consommateurs, mais sans pénaliser les acteurs respectueux de la loi. Mieux protéger les consommateurs contre la fraude et contre les abus, c'est très concret. C'est, par exemple, encadrer les obligations de transparence du démarcheur au début de la conversation engagée avec le consommateur. C'est aussi limiter les cas de démarchage légitime, et je voudrais ici revenir sur l'article 5, qui a été supprimé par la commission des lois ; je rappelle tout de même son but : exiger un lien direct entre le démarchage et les contrats en cours. On ne peut pas vous appeler pour des produits qui n'ont aucun rapport avec les contrats que vous possédez. Nous aurons de nouveau ce débat, mais le Gouvernement défendra fermement le rétablissement de cet article qui me paraît important pour les consommateurs. consommateurs. Nous ne devons pas nous tromper de cible. La cible, ce sont les fraudeurs, et non le démarchage téléphonique en tant que tel. Le Gouvernement est donc très réservé sur tout ce qui peut pénaliser le démarchage respectueux de la réglementation derrière ces mesures qui ne sont pas toujours efficaces contre la fraude. Par ailleurs, il y a parfois une vraie menace pour les TPE et les PME, et pour de nombreux emplois. Il ne s'agit pas de n'importe quels emplois les centres d'appel sont souvent un premier accès à l'emploi pour des publics fragiles ; ces emplois sont flexibles et permettent d'apporter un complément de revenu à des personnes qui ne peuvent pas travailler à temps plein- je pense notamment aux mères célibataires. C'est cette réalité économique et sociale qui nous interdit de soutenir certaines mesures radicales comme un systématique. Je traduis en bon français : c'est partir du principe que le consommateur est toujours contre le démarchage et donc interdire celui-ci, sauf demande explicite du client. Si l'on veut tuer tout ce secteur d'activité, on le peut ; mais tel n'est pas notre but. Alors, comment lutter efficacement contre la fraude et le harcèlement ? La meilleure solution, c'est d'abord de renforcer Bloctel. Il faut que ce dispositif soit mieux connu et que son contournement soit plus sévèrement sanctionné. Nous sommes favorables au renforcement des sanctions à l'égard des entreprises qui pratiquent le démarchage téléphonique sans soumettre leur liste à Bloctel pour que ces sanctions soient réellement dissuasives. À ce jour, plus de cent procès-verbaux administratifs ont été dressés et trois procédures pénales engagées. Il faut aussi sensibiliser les consommateurs à l'importance des signalements et à la nécessité de bien renseigner Bloctel au sujet des appels reçus. Cela fera l'objet d'une action de communication, qui sera également dirigée vers les entreprises ; à ce jour, environ sept cents entreprises ont adhéré à Bloctel, ce qui est très insuffisant. Enfin, l'interface de Bloctel doit être évaluée et améliorée. Il nous faut aussi lutter contre les autres pratiques frauduleuses qui occasionnent des appels intempestifs

appels émanent très souvent de professionnels établis à l'étranger. C'est pourquoi, là encore, les consommateurs doivent être mieux informés des mesures prises pour les protéger. Nous venons de rendre obligatoire l'offre, par les opérateurs téléphoniques, d'une option de blocage des appels des abonnés vers les numéros surtaxés.

politique traite bien du démarchage téléphonique, qu'elle est proportionnée, et qu'elle laisse à l'administration l'appréciation d'un droit à l'erreur pour les TPE et les PME, le Gouvernement y est favorable. Elle dissuadera fortement les entreprises, je n'en doute pas. sont les brefs messages que je tenais à vous présenter. Nous sommes déterminés à identifier toutes les pistes envisageables pour mieux réguler le démarchage, faire cesser ces nuisances et sanctionner les fraudes. Toutefois,

madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, que nous examinons aujourd'hui, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 6 décembre dernier. Elle était présentée par notre collègue député Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues. Le démarchage téléphonique, ou prospection commerciale, se définit comme la prise de contact par téléphone avec un consommateur

le consentement préalable du consommateur à faire l'objet de prospection commerciale n'étant pas exigé. Depuis 2014, un dispositif législatif permet aux consommateurs de faire valoir leur opposition aux démarchages téléphoniques, par l'inscription au service Bloctel. Il est alors interdit à un professionnel de démarcher un consommateur qui se serait inscrit sur cette liste. Tout manquement est passible de sanctions administratives, lesquelles ne peuvent excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Plusieurs exceptions à ce principe sont prévues, notamment en cas de relations contractuelles préexistantes entre le professionnel et le consommateur, ainsi que pour la presse, pour les activités des associations à but non lucratif ou pour les instituts de sondages. La gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel, est assurée par Opposetel, le délégataire de service public désigné pour cinq ans, la délégation prenant fin en 2021.

Le nouveau règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, applicable depuis mai dernier, ne remet d'ailleurs pas en cause la possibilité pour les États d'opter pour un système d'opposition en matière de démarchage téléphonique. Le droit de l'Union européenne n'impose en effet le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée- courriels, SMS, télécopies.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation ; pêle-mêle : le non-respect par certaines entreprises de leur obligation réglementaire de mise en conformité de leurs fichiers-

De même, la recrudescence des pratiques frauduleuses qui ne rentrent pas dans le champ du démarchage téléphonique, mais qui sont perçues comme telles par les consommateurs, tend à renforcer le mécontentement

sans déstabiliser le secteur du démarchage téléphonique, d'où cette notion d'équilibre, soulignée par Mme la secrétaire d'État. L'article 1 de la proposition de loi consacre dans la loi l'obligation pour tout professionnel de faire vérifier ses fichiers de prospection par l'organisme à qui est confiée la gestion de Bloctel. La méconnaissance de cette obligation serait passible d'une amende dont le montant serait par ailleurs considérablement renforcé. Tout en approuvant ce principe, qui vise à répondre à l'une des insuffisances du système actuel, la commission a précisé les modalités de vérification des fichiers de prospection commerciale en cas de sous-traitance. De même, elle a approuvé le renforcement des sanctions administratives en cas de manquement des professionnels à la législation relative au démarchage téléphonique, et la publicité donnée à certaines sanctions. Elle a toutefois encadré le régime des sanctions administratives en cas de manquements simultanés à plusieurs obligations, ou de cumul avec une sanction pénale, afin d'en assurer la proportionnalité, compte tenu de l'augmentation du montant des amendes susceptibles d'être prononcées. Celles-ci pourraient en effet désormais atteindre 375 000 euros pour une personne morale, contre 75 000 euros

ou pénales ; je le regrette, je m'en expliquerai tout à l'heure, vous le comprendrez. La commission s'est également opposée à la limitation de « l'exception client », par laquelle un professionnel peut contacter un consommateur même s'il est inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique- c'est le fameux article 5 du texte -, et a souhaité maintenir le droit en vigueur qui permet au professionnel de contacter un consommateur avec lequel il a des « relations contractuelles préexistantes », ce qui doit être interprété comme concernant

des emplois sont en jeu, chacun doit l'avoir présent à l'esprit. La commission a aussi renforcé la transparence et la déontologie du secteur du démarchage téléphonique, en prévoyant le respect de normes déontologiques, et en créant un régime de données ouvertes, ou, applicable à l'organisme gestionnaire du service Bloctel, de façon à mieux contrôler son activité. Je sais que le Gouvernement y est défavorable ; cela m'étonne beaucoup. Nous y reviendrons, madame la secrétaire La commission des lois s'est enfin montrée favorable à la philosophie des articles 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à lutter contre les pratiques frauduleuses, celles-ci représentant une grande partie des nuisances subies par les consommateurs. L'article 6 définit notamment les conditions dans lesquelles les opérateurs exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée doivent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux. La commission a conforté la sécurité juridique de ces outils. Le Gouvernement propose de supprimer l'une des précisions que nous avons apportées concernant la certification des signalements des consommateurs ayant relevé des anomalies sur des numéros surtaxés, dans des conditions définies par voie réglementaire, au motif d'une absence de souplesse du dispositif. Je n'ai pas de religion en la matière, madame la secrétaire d'État, mais je n'estime pas forcément opportun de supprimer tout principe de certification ou de s'en remettre uniquement à l'autorégulation des opérateurs

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'encadrement, voire la limitation stricte, du démarchage téléphonique est un véritable serpent de mer de la protection des consommateurs. En 2011, déjà, le groupe du RDSE avait présenté et fait adopter par le Sénat une proposition de loi, plus ambitieuse que celle-ci, qui prévoyait le passage de l'à l', c'est-à-dire à l'obligation de recueillir le consentement préalable du consommateur, en amont de toute activité de démarchage par voie téléphonique. À l'époque, Jacques Mézard avait résolument dénoncé les dérives constatées dans ce secteur d'activité, qui confinent parfois au harcèlement des consommateurs. Ces dérives touchent particulièrement les personnes âgées ou vulnérables, et celles qui utilisent encore le téléphone fixe, dont l'usage, en raison des évolutions technologiques, se fait de plus en plus rare.

Face à ces pratiques commerciales agressives, de nombreuses sociétés de télémarketing n'hésitant pas à appeler les personnes plusieurs fois dans le même mois, à des horaires inopportuns, en soirée ou le week-end, il paraît en effet indispensable de renforcer les droits des citoyens. Ceux-ci devraient pouvoir ne plus être importunés chez eux et assaillis d'offres et d'informations commerciales diverses qu'ils n'ont pas sollicitées. On peut donc regretter que la proposition de loi de 2011 n'ait jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Une autre proposition de loi, présentée l'an dernier par le député Pierre Cordier, reprenait le principe de l'. Elle a été adoptée par les députés, mais après la suppression de son article 1, qui en portait le dispositif principal ; autant dire qu'elle a été vidée de sa substance ... Puisque l'on parle de serpent de mer, je pense aussi au sujet connexe de la localisation des centres d'appel, secteur évalué à plus de 250 000 emplois en France. Le rapport du député Marc Le Fur de 2012 indiquait qu'une grande partie des centres d'appel était néanmoins située à l'étranger, principalement dans des pays francophones à bas coûts- le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal -, mais également dans des pays européens- Portugal ou Roumanie.

succès. On invoque souvent le fait que les plateformes sont situées à l'étranger pour expliquer les entorses au droit français, mais les textes européens sur le conflit de lois sont clairs relatifs à la consommation sont en principe régis par la loi du pays de résidence habituelle du consommateur. Cela semble logique dans la mesure où c'est la loi de ce pays qui prévoit le niveau de protection auquel le consommateur peut légitimement s'attendre, et ce, même si le professionnel n'exerce pas son activité dans l'Union européenne. Enfin, plusieurs de nos partenaires européens ont d'ores et déjà opté pour le régime du consentement préalable- l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Danemark -, ce qui montre que le changement de régime n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, la présente proposition de loi devrait rencontrer un meilleur succès que les tentatives passées. Il est vrai que son approche est différente, d'aucuns diront « plus timide », dans la mesure où elle conserve le régime actuel de la désinscription, tout en tentant de le rendre plus efficace. dit, son objet est plus large, puisqu'elle concerne aussi la lutte contre les appels frauduleux, ce à quoi l'on ne peut que souscrire. Je salue certains apports de la commission concernant, par exemple, les informations à délivrer obligatoirement au consommateur lors d'un démarchage, ou encore l'accessibilité des données essentielles de l'organisme gérant la liste d'opposition. En revanche, pourquoi avoir supprimé l'article 5 qui encadrait davantage l'exception client, c'est-à-dire la possibilité de démarchage lorsque des relations contractuelles préexistent ? Pour le reste, la commission a conservé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, aggravant notamment fortement les sanctions en cas de manquement à diverses dispositions relatives aux professionnels, de décliner son identité et la nature commerciale de son activité, l'interdiction de recourir aux numéros masqués ou encore la nécessité de vérifier régulièrement la liste d'opposition. On passe ainsi à des sanctions vingt-cinq fois plus sévères. Les mesures de lutte contre les pratiques frauduleuses- rappel à un numéro surtaxé sans offre réelle, appels en absence, SMS frauduleux, et j'en passe -vont aussi globalement dans le bon sens. c'est mon dernier point -, les solutions ne relèvent pas uniquement, ni peut-être essentiellement, du domaine de la loi. Elles doivent passer par un renforcement des contrôles opérés par la DGCCRF, dont les agents sont habilités à rechercher et à constater les manquements au cadre régissant l'opposition au démarchage téléphonique. Ces contrôles sont aujourd'hui insuffisants. Une autre piste, évoquée par le rapporteur, est la réduction du coût d'utilisation du service de vérification des listes d'opposition pour les entreprises et, surtout, l'amélioration du fonctionnement du service d'opposition Bloctel, dont les résultats sont pour l'instant très décevants. Enfin, plus généralement, il faut améliorer la connaissance par les entreprises de leurs obligations et par les consommateurs de leur droit

Les amendements de ma collègue Nathalie Delattre, que je défendrai tout à l'heure, portant sur la mise en place d'un préfixe et sur l'encadrement des dates et horaires de démarchage vont dans ce sens. Pour le reste, conscients des enjeux tant en termes d'emploi que de droit au respect de la vie privée et à la tranquillité, nous déterminerons notre vote à l'issue des débats.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes heureux que le Sénat examine cette proposition de loi qui vise à mieux protéger les droits des consommateurs face au démarchage téléphonique intempestif ou frauduleux. En effet, ces appels représentent trop souvent une nuisance pour nos concitoyens ; les premières victimes de ces pratiques intrusives sont les personnes les plus présentes à leur domicile : des jeunes, voire des très jeunes, ou des personnes âgées, autrement dit, des personnes plus vulnérables.

Malheureusement, il n'en est rien ; ce dispositif, qui présente aujourd'hui de graves lacunes, requiert de profondes améliorations. C'est la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, qui a mis en place cette liste Bloctel, dans le but d'offrir aux consommateurs ne souhaitant plus faire l'objet de démarchage téléphonique la possibilité de s'y enregistrer.

ou a très peu baissé. Le constat est donc sans appel : le cadre actuel ne permet pas à cet outil d'être efficace. C'est pourquoi nous voulons tout d'abord saluer le travail de notre collègue député Christophe Naegelen, qui a déposé ce texte équilibré, ô combien nécessaire, que l'Assemblée nationale a adopté le 6 décembre dernier à l'unanimité. de loi que nous examinons aujourd'hui est fondée sur une logique d'- désolé pour cet anglicisme -, qui offre un droit d'opposition, à condition de s'être inscrit sur la fameuse liste Bloctel. Cette approche s'oppose au système d', qui exige un consentement exprès et exprès et préalable au démarchage. Ce dernier système, séduisant au premier abord, pourrait avoir des effets contre-productifs. Aussi, comme notre commission des lois, nous souhaitons conserver le système d', qui qui permet, lorsqu'il est bien encadré, d'offrir un moyen simple de contrecarrer ce harcèlement téléphonique, sans pour autant détruire une activité économique qui représente, selon les chiffres de notre rapporteur, près de 56 000 emplois en France. premier lieu, il est essentiel d'obliger les démarcheurs à décliner clairement leur identité, l'objet de leur appel, mais aussi à informer chaque individu de la possibilité de souscrire à la liste d'opposition. En second lieu, la question des sanctions financières est cruciale pour s'opposer à la pugnacité des entreprises de démarchage. Les sanctions plus élevées prévues par ce texte devraient enfin- nous l'espérons -permettre de les dissuader d'enfreindre les règles. Nous avons eu la surprise de voir disparaître l'article 5 du texte en commission nous persistons à penser que, lorsqu'une personne est inscrite sur Bloctel, l'exception permettant malgré cela de la solliciter doit être strictement encadrée. En effet, le droit en vigueur dispose qu'un consommateur ayant des relations contractuelles préexistantes avec un professionnel peut être démarché par celui-ci, même s'il est inscrit sur Bloctel. de l'article 5, l'Assemblée nationale a restreint le périmètre concerné, en proposant que seules les sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours puissent donner lieu à un démarchage. Nous soutenons cette rédaction, et je vous proposerai donc un amendement tendant à la rétablir. Ce texte a identifié les lacunes du cadre actuel, et il tente d'y répondre de manière concrète. Face à l'agacement légitime des Français, face à des professionnels du démarchage souvent peu scrupuleux, nous devons agir rapidement.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

ou à ce que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. Il s'agit d'un mécanisme où le consentement est supposé acquis, mais où la liberté est laissée aux consommateurs de refuser le démarchage.

Les consommateurs peuvent ainsi s'inscrire sur une liste répertoriant les personnes ne souhaitant pas être démarchées, liste que doivent consulter les entreprises avant toute opération. Or, si le fichier Bloctel a permis d'obtenir certains résultats significatifs, plusieurs lacunes viennent en altérer l'efficacité. Tout d'abord, le nombre d'entreprises qui soumettent leurs fichiers à Bloctel, pour les expurger des données téléphoniques des particuliers inscrits, est trop faible. Ensuite, l'autorité administrative, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, organise trop peu de contrôles, et ceux-ci conduisent à trop peu de sanctions.

De plus, ces sanctions ne sont jamais publiées, elles n'ont donc aucun effet sur l'image de marque d'une société, ce qui- vous en conviendrez -en atténue grandement la portée. À côté des démarchages commerciaux intempestifs et illégaux, les Français subissent aussi, de plus en plus fréquemment, des pratiques frauduleuses fondées sur des numéros surtaxés. Ces pratiques touchent particulièrement les publics les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les adolescents, appâtés par la promesse de places de spectacle, de produits de mode ou de gains d'argent.

consiste à inciter les consommateurs à composer, pour des raisons trompeuses, ces numéros dits de « service à valeur ajoutée », et à les pousser à multiplier les appels ou à rester le plus longtemps possible en ligne. ligne. Cette proposition de loi répond donc à un double objectif. D'une part, elle vise à renforcer l'effectivité du droit d'opposition au démarchage téléphonique ; d'autre part, elle tend à mieux lutter contre la fraude.

l'incitation à la mise en place d'un code de déontologie et de la création d'un régime de données ouvertes, applicable à l'organisme gestionnaire du service Bloctel, de façon à mieux contrôler son activité. Je me félicite également qu'elle ait précisé les modalités de vérification des fichiers de prospection commerciale en cas de sous-traitance. Enfin, parmi les modifications apportées, je veux souligner particulièrement celle qui conforte la sécurité juridique des outils permettant de lutter contre les pratiques frauduleuses, qui représentent une grande partie des nuisances subies par les consommateurs, notamment en subordonnant toute résiliation de contrat d'un éditeur de numéro surtaxé frauduleux à une mise en demeure infructueuse. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je partage sans réserve l'esprit de ce texte qui entend défendre les droits de nos concitoyens. En effet, la question du démarchage téléphonique abusif ou frauduleux nous concerne tous.

la tentative d'effraction dans l'espace privé au moyen du démarchage téléphonique est un authentique fléau, dont, hélas, le remède thérapeutique nous échappe encore. quand bien même nous le trouverions, il n'est pas certain que l'exaspération de nos citoyens en ressortirait diminuée, tant on observe, chiffres à l'appui- ils ont été cités précédemment -, la recrudescence de pratiques frauduleuses qui n'entrent pas dans le champ du démarchage téléphonique, fussent-elles fussent-elles perçues comme telles par les consommateurs qui en subissent le préjudice. Ces pratiques consistent, dans leur forme majoritaire, à inciter le consommateur à appeler un numéro surtaxé, sans qu'aucun produit ou service réel soit, en contrepartie, mis à sa disposition.

à défaut d'éliminer la chose, nous inventons le mot censé nous en préserver ... Pourtant, rien n'y fait, ce fléau n'en finit pas ; les Français s'en agacent, et, sur ce terrain, le législateur paraissait bien désarmé. Nos débats illustrent ces tribulations. La prospection téléphonique intempestive a été rebattue sous toutes ses coutures : d'abord à l'Assemblée nationale, puis par notre honorable commission, sans toutefois que nous parvenions à soulager notre scepticisme quant à l'apport réel de l'ouvrage législatif. À notre décharge, l'opérationnalité du système de consentement préalable, dit, ne relève pas uniquement du périmètre de la loi. périmètre de la loi. Toutefois, sans revenir sur la philosophie générale de ce principe, on mesure combien il peut être hasardeux de légiférer sur un mécanisme protectionniste sous l'effet duquel toute une économie souterraine de prospection commerciale frauduleuse menace de prospérer. Ainsi donc, et quoi qu'on en pense par ailleurs, cette entreprise de régulation n'est pas une mince affaire. Bien évidemment, il ne faut pas renoncer. La ligne de crête est étroite entre le spectre de la délocalisation salariale- contrepartie logique du système de non-consentement préalable -et un nécessaire protectionnisme à l'attention des consommateurs désabusés. Notre commission avait à coeur d'établir un point d'équilibre acceptable entre, d'une part, cette protection accrue des consommateurs et, d'autre part, le maintien sur le territoire national d'une activité économique pourvoyant un nombre non négligeable d'emplois, dans le strict respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie. Elle a mené un remaniement rédactionnel.

Nous nourrissons quelques soupçons quant au caractère opérationnel de dispositions législatives dépourvues, à ce stade, d'étude d'impact préalable. En lieu et place serait prévue une mise à disposition en, par la société Opposetel, des « données essentielles » de son activité, qui seront également transmises au Conseil national de la consommation. Ce dispositif nous semble insuffisant pour dresser un diagnostic précis du fonctionnement de la liste d'opposition et de sa gouvernance. La commission a retenu une juste proportionnalité du régime des sanctions administratives en cas de manquements simultanés à plusieurs obligations ou de cumul avec une sanction pénale à l'article 3. Cette logique généralisante fait pourtant peu de cas, semble-t-il, du principe de proportionnalité dont elle se réclame nous priverions ainsi l'autorité administrative compétente de la possibilité de prononcer des amendes d'un montant adapté à la gravité des manquements constatés. nous craignons le caractère rigide et désincitatif du dispositif de certification des signalements par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'article 6. Nous sommes pleinement favorables à la limitation de « l'exception client

Notre groupe aurait apprécié un vote conforme, la prochaine niche UDI n'intervenant qu'en décembre prochain. Cette prolongation de la navette sera toutefois utile pour prendre connaissance des consultations engagées auprès des associations de consommateurs. Comme vous l'aurez compris, mes chers collègues, si nous

des numéros surtaxés et à améliorer le fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage, dite Bloctel. Les mots ont un sens. Parlez aujourd'hui de démarchage téléphonique et on vous répondra, selon les cas

en effet restées « au milieu du gué », laissant les citoyens seuls face à cette plaie qu'une simple interdiction suffirait à éradiquer. Si on connaît le poids des lobbies, on ne reste pas moins dubitatif devant un tel manque de volonté face à une activité une activité économique dont le caractère indispensable ne saute pas aux yeux. La publicité et la suggestion perpétuelle à la consommation ont envahi nos vies comme jamais dans notre histoire : sur les murs de nos villes, que la loi de 1881 interdit pourtant à l'expression des citoyens,

citoyen, dans l'intimité, se retrouvait libre de se dégager de ces incitations publicitaires en éteignant la télé, en choisissant quel journal acheter, en changeant de station de radio ... Or le démarchage téléphonique a la particularité de s'attaquer au dernier rempart, à la dernière zone libre de réclames : l'intimité domestique.

Ce principe de consentement préalable est le seul qui permette de garantir une protection des consommateurs. J'entends bien les arguments concernant les emplois qui pourraient être menacés ou la difficulté dans laquelle seraient plongées certaines sociétés vivant de ces activités. Allons au fond des choses et du débat. De quoi parlons-nous ? De défense des emplois ou des profits ? S'il s'agit de préserver les emplois, commençons par rapatrier ceux qui sont délocalisés à l'étranger, dans des pays francophones à plus bas salaires,

ou si peu au développement de leur propre société ? C'est un autre type de coopération qu'il convient de mettre en oeuvre. Intéressons-nous également aux conditions de travail et au niveau des rémunérations dans les centres d'appels sur notre territoire. Posons-nous la question de l'utilité sociale de ce secteur économique. N'y a-t-il pas mieux à faire, n'y a-t-il pas plus utile que de déranger les gens dans leur vie quotidienne, à n'importe quelle heure, pour vendre tout et n'importe quoi ? Pourquoi ne pas « réinventer » ces emplois ? Nos concitoyens souffrent- ils nous le disent aujourd'hui -d'une profonde déshumanisation, d'un vide où le téléphone ou internet sont censés remplacer l'humain. Je ne m'éloigne pas du sujet en rappelant que les centres d'appels, comme les plateformes numériques, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, par économie d'emplois et par profits, participent aussi d'une profonde déstructuration de notre société et d'une désertification de nos territoires. Redonnons du lien social, du sens à la société. Privilégions les rapports humains, que ce soit dans l'activité commerciale, dans l'après-vente, dans l'accès aux services publics ou aux organismes sociaux. Nous pouvons transformer ces emplois en emplois utiles socialement et économiquement, derrière un téléphone et derrière un guichet, au réel service des usagers et des consommateurs citoyens. Le texte qui nous est présenté n'est pas, de notre point de vue, à la hauteur de ces enjeux.

nécessaire. La responsabilité accrue donnée aux opérateurs de téléphonie souligne ce manque d'ambition de l'État concernant ses instances de contrôle et marque le défaussement de ses prérogatives sur des opérateurs privés qu'aucune instance démocratique ne contrôle et et qui se voient offrir de plus en plus de pouvoir. Au-delà de toutes les critiques, positives ou négatives, que nous pourrions émettre sur ce texte, notre groupe tient à rappeler sa volonté d'inverser le dispositif

le développement du capitalisme étant ce qu'il est, la loi de la marchandise allait s'étendre sur le monde réel, concret. Quand on voit les entrées de ville avec ces univers de pancartes, de parallélépipèdes en tout genre, on comprend que la loi de la marchandise a pris possession de l'espace.

par des quantités de démarches téléphoniques, à toutes les heures, tout simplement parce qu'il faut vendre et parce que la loi de la marchandise s'inscrit dans le temps de la vie quotidienne comme elle s'inscrit dans son espace. Nous en Nous en avons véritablement l'illustration avec ces quantités de coups de téléphone qui finissent par exaspérer nos concitoyens.

qui permet aux citoyens de s'inscrire gratuitement sur une liste officielle pour exprimer leur refus du démarchage téléphonique. Cette loi pose une double interdiction aux entreprises : d'une part, l'interdiction de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel pour son compte, un consommateur inscrit sur cette liste, sous peine d'une amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes part, l'interdiction de céder à un tiers, qu'il s'agisse de location ou de vente, des fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou de plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

positif. Ce choix nous paraît tout à fait réaliste. Il permet de répondre au fléau que représente ce démarchage non sollicité et à l'efficacité toute relative du dispositif Bloctel. Il s'agit d'aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et des courriels, comme on dit aussi en français, qui repose sur un système d'accord express du consommateur afin de s'assurer que seules les personnes qui se sont inscrites volontairement seront démarchées. Il s'agit aussi de mieux encadrer l'exception prévue à l'article L. 223-1

Deuxièmement, il faut, nous semble-t-il, s'inscrire dans la continuité du nouveau règlement général européen de protection des données personnelles, dit RGPD, qui a fait l'objet d'un projet de loi visant visant à l'adaptation du droit national, adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 14 mai 2018. Troisièmement, cet encadrement est aussi souhaité par un nombre non négligeable d'entreprises, celles qui démarchent ou prospectent d'une manière honnête, contrôlée et légitime. Les professionnels des centres d'appels soulignent eux-mêmes que les appels intempestifs portent atteinte à tout le monde, mais portent aussi préjudice au démarchage classique et justifié. D'une certaine façon, les mauvais appels tuent les bons,

un identifiant d'appel obligatoire, qui permettrait d'informer le consommateur de la nature de l'appel avant de décrocher. Il devrait être possible de mettre un tel dispositif en place. Enfin,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la lutte contre le démarchage téléphonique intempestif et contre les appels frauduleux apparaît comme nécessaire pour un grand nombre de consommateurs. Qui n'a jamais songé à débrancher son téléphone fixe dans le seul but d'éviter le démarchage intempestif d'entreprises souhaitant vendre, qui de nouvelles fenêtres, qui des panneaux solaires, quand bien même ces achats seraient inutiles ? Qui ne s'est jamais senti excédé de recevoir de faux messages invitant à passer un coup de téléphone à un numéro finalement frauduleux ? Sans doute connaissez-vous des proches qui n'ont plus de téléphone fixe pour éviter ces appels intempestifs et intrusifs, majoritairement passés à des heures où les familles sont réunies, le midi, ou après les heures de travail. Il a en effet été constaté que le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés peuvent avoir un pouvoir de nuisance considérable sur l'ensemble de notre population et de notre économie. On considère que près de 40 % des appels intempestifs faisant l'objet de signalements des consommateurs ne relèvent pas du démarchage légal, mais bien d'un appel frauduleux. Plusieurs pratiques de fraude sont mises en place pour flouer le consommateur. La première consiste à appeler un numéro de téléphone en ne le laissant sonner qu'une fois. La personne appelée, qui n'a pas réussi à décrocher à temps, essaie généralement de rappeler le numéro en question.

Une autre technique de fraude consiste à appeler un consommateur en lui indiquant qu'il doit rappeler un numéro, lui aussi surtaxé, pour réceptionner un colis, demander un rendez-vous médical ou autre- l'imagination des arnaqueurs est sans limite Lorsque le consommateur rappelle ce numéro, sans savoir s'il s'agit d'une arnaque ou pas, il est généralement gardé au bout du fil le plus longtemps possible par le téléopérateur, qui ne lui indique que très rarement que le numéro est surtaxé. Bien des victimes se rendent compte de l'arnaque lorsqu'elles reçoivent leur facture de téléphone et doivent s'acquitter, hors forfait, de sommes considérables. Une variante de ce procédé consiste à organiser des appels par le biais de robots qui laissent des messages vocaux au consommateur pour l'inciter à rappeler son banquier ou son médecin, par exemple, par le biais d'un numéro également surtaxé. Les mécanismes de micropaiement par téléphone sont aussi une source inépuisable d'abus de faiblesse. Ne requérant pas d'accord parental, ils exposent particulièrement les enfants et les adolescents. Toutes ces pratiques frauduleuses reposent sur une usurpation de numéro de téléphone permettant aux fraudeurs de réduire leur traçabilité par les pouvoirs publics.

Ces pratiques trompeuses, qui peuvent s'apparenter à du harcèlement téléphonique, voire à des abus de faiblesse, sont majoritairement mises en place contre nos populations les plus vulnérables. Les enfants, les adolescents, mais aussi les chômeurs ou les retraités sont généralement moins armés pour lutter contre la pression à l'achat. Chaque année, 40 000 de nos aînés sont victimes d'abus de faiblesse. Certains, Certains, conscients qu'ils sont les cibles privilégiées d'entreprises ou d'acteurs peu scrupuleux, ne daignent même plus répondre sur leur téléphone fixe, ce qui peut parfois mettre leur santé en danger, leurs proches ou leurs soignants essayant de les joindre sans succès. Chez nos concitoyens les plus vulnérables, davantage présents à leur domicile, ce démarchage intempestif se nourrit de leur vulnérabilité pour leur faire acheter des biens majoritairement inutiles des panneaux solaires, alors qu'ils vivent en appartement, des assurances qui ne s'appliquent pas à leur situation, ou même des gadgets qui contribuent, dans les cas les plus sérieux, à aggraver un surendettement chronique.

Les faibles perspectives de remboursement contribuent à empirer ce sentiment d'impuissance des consommateurs floués. Un constat est donc très largement partagé, tant par les consommateurs que les parlementaires

entre une protection renforcée des consommateurs et le maintien, sur le territoire national, d'une activité économique d'importance. Je voterai donc en faveur de cette proposition de loi de cette proposition de loi en gardant toujours à l'esprit qu'il nous faudra rester particulièrement vigilants, les fraudeurs redoublant systématiquement d'imagination pour contourner la réglementation et nuire à nos concitoyens. La parole est

le cadre actuel de protection des consommateurs face au démarchage téléphonique n'est pas efficace et ne protège pas suffisamment leurs droits au quotidien. Après le constat de ces lacunes, partagé sur toutes les travées de notre hémicycle, vient le temps des réponses. Le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui

Nous pourrions aller plus loin, il est vrai. Nous préférons aujourd'hui conserver l'esprit du texte voté à l'Assemblée nationale, dont je salue la grande qualité. Comme le président Hervé Marseille, je tiens également à saluer le travail de notre collègue député Christophe Naegelen.

renforcées et une responsabilisation accrue des opérateurs. Comme Hervé Marseille, je regrette la remise en cause de l'article 5 du texte, qui, je le rappelle, prévoyait une exception de taille au service Bloctel. C'est assurément un mauvais signal envoyé à nos concitoyens et un renoncement incompréhensible. Il faut garantir aux citoyens inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique des sollicitations minimes qui se justifient uniquement par un contrat en cours. Face à

tranquillement chez vous, en famille, à l'heure du dîner ou du déjeuner, quand soudain le téléphone sonne ... Au bout du fil, un étudiant ou un téléopérateur vous appelle le plus souvent depuis une plateforme localisée au Maghreb pour

Soyons honnêtes, cette situation ne convient à personne. Il est urgent de protéger nos concitoyens en améliorant le cadre législatif. Le démarchage téléphonique est une plaie- c'est bien ainsi que le ressentent les Français. L'enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir en 2017 montrait que toutes les personnes y ayant répondu jugeaient le démarchage téléphonique « agaçant 92 % d'entre elles « trop fréquent ». Selon le sentiment général, il ne cesse d'augmenter. Au-delà de la gêne que constitue cette pratique, il n'est pas rare, comme le montrent les rapports de mes collègues André Reichardt et Christophe Naegelen, député, de constater une véritable pression à l'achat, voire un abus de faiblesse, notamment sur des publics vulnérables comme les jeunes adolescents ou les personnes âgées. Nombreux sont ceux qui sont victimes d'arnaques, organisées par des sociétés ne proposant aucun service à valeur ajoutée, appelant en des numéros surtaxés, demandant l'envoi de SMS pour récupérer des codes qui ne donnent accès à rien

C'est absolument considérable ! L'article 6, tel qu'il était prévu dans le texte original déposé à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2018 par le député Naegelen et plusieurs de ses collègues, prévoyait, dans son avant-dernier alinéa, que les sommes liées à ces surtaxes frauduleuses seraient utilisées dans un premier temps pour le financement d'un outil permettant aux opérateurs de réaliser un suivi et de rembourser le consommateur. Une fois cet outil développé, les sommes en question leur auraient été effectivement rendues. Je regrette beaucoup que cette disposition permettant le remboursement des consommateurs escroqués ait été supprimée par l'amendement déposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée J'entends bien l'argument selon lequel l'intervention n'aurait pas été légale, dans la mesure où le blocage des reversements ne peut être imposé en l'absence de décision judiciaire. Néanmoins, il aurait été souhaitable de trouver une solution permettant le remboursement des consommateurs,

Comprenez le sentiment d'injustice terrible des consommateurs escroqués, surtout eu égard aux immenses bénéfices de ces pratiques frauduleuses ! Je regrette également que l'article 5 ait été supprimé en commission. Il prévoyait que les professionnels ne pouvaient démarcher des clients que pour des biens et services ayant un rapport direct avec l'objet du contrat en cours, et non plus pour ceux liés à des relations contractuelles préexistantes. Il a été invoqué le fait que cette décision mettrait en difficulté un certain nombre d'entreprises, dont le démarchage est essentiel au développement, voire à la survie. C'est la raison pour laquelle a été écartée l'idée d'instaurer un consentement préalable au démarchage, en considérant ces appels interdits, sauf à donner l'autorisation d'être démarché.

La disposition restreignant les appels des démarcheurs à ceux ayant un rapport direct avec l'objet du contrat en cours ne me paraissait pas exagérée. protéger les emplois liés à cette activité, qui sont au nombre de 50 000 en France, mais il serait bon aussi de se donner les moyens de répondre aux attentes de nos compatriotes, en bannissant des pratiques qui s'apparentent au harcèlement.

L'esprit de cette proposition de loi doit rester la protection des consommateurs. Dès lors, même s'il faut éviter de fragiliser notre tissu économique, on ne peut pousser son développement en encourageant le démarchage des personnes, en particulier des personnes vulnérables. Téléphone, téléphonie mobile, télévision, internet, tous ces moyens de communication ont envahi notre quotidien. Dans ces conditions, ils deviennent des instruments économiques, commerciaux et des moteurs du développement. Le démarchage téléphonique est aujourd'hui devenu une pratique courante. Il s'est développé de manière exponentielle et, il faut le dire, souvent anarchique,

Nous considérons en effet que le dispositif Bloctel est insuffisant, voire inefficace, car il suppose une démarche volontaire du consommateur,

liste. À nos yeux, tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est à son domicile. Seuls les consommateurs acceptant d'être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition. Cet amendement vise tout simplement à prévoir le consentement préalable, positif et exclusif.

La parole est à M. Antoine Lefèvre. Cet amendement, que je présente au nom de Mme Corinne Imbert et qui a été cosigné par un grand nombre de collègues, vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus par son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché. Cet amendement vise à limiter le démarchage abusif, intempestif et, surtout, non sollicité.

il semble indispensable, pour renforcer sa protection, que le numéro qui s'affiche lors d'un appel soit précédé d'un identifiant d'appel, afin qu'il soit informé en amont de la nature de l'appel et puisse, le cas échéant, décider ou non de décrocher. Depuis la loi de 2014 relative à la consommation, l'appel doit être affecté à l'entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut s'agir du numéro du centre d'appels, qui peut être situé à l'étranger, ou du numéro d'une autre entreprise. Par ailleurs, l'article L. 221-17 du code de la consommation ne mentionne pas l'obligation d'utiliser un indicatif unique. Les numéros employés par les démarcheurs sont ainsi multiples et non identifiables par les consommateurs. En outre, cette absence d'indicatif unique ne permet pas de lutter contre des pratiques frauduleuses telles que l'usurpation de numéro. Les sociétés pratiquant le démarchage téléphonique n'ont plus le droit de passer des appels en numéro masqué et le numéro qu'elles affichent doit permettre de rappeler le prestataire du produit, et non le centre d'appels. Or certaines entreprises parviennent à afficher sur le téléphone du destinataire un autre numéro que le leur, afin de ne pas être identifiées ou de cacher le fait qu'elles appellent de l'étranger. Cette technique, appelée

empêcherait les démarcheurs téléphoniques de contourner certaines dispositions légales, ainsi que les dispositifs physiques d'opposition au démarchage, et garantirait une meilleure identification du démarchage par les particuliers. Cette proposition va dans le sens d'une plus grande protection du consommateur.

Si le droit interdit déjà aux démarcheurs d'utiliser des numéros masqués, l'affichage actuel des numéros n'apparaît pas satisfaisant au regard des enjeux de transparence et de protection des consommateurs portés par la présente proposition de loi. C'est pourquoi cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d'appel obligatoire, qui permettra d'informer le consommateur de la nature de l'appel avant de décrocher. L'instauration d'un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l'encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l'appel. Elle permettra en particulier de savoir s'il s'agit d'un appel à caractère commercial. À défaut de l'adoption de cet amendement, une étude de faisabilité, qui a été évoquée en commission des lois, paraît plus que souhaitable. Les deux amendements

L'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique n'est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu'un système concernant les appels téléphoniques permette une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il serait possible d'imaginer un système de serveur vocal interactif.

pour faire simple et en bon français, monsieur Sueur, d'. Ils tendent ainsi à revenir sur le système actuel fondé sur l'opposition expresse du consommateur au démarchage téléphonique. Le système de l', quelle que soit sa forme- consentement préalable du consommateur lors de la souscription d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou consentement préalable exprès auprès de chaque entreprise qui en ferait la demande au consommateur -reviendrait à une quasi-interdiction de l'activité des centres d'appels.

démarchés au téléphone ? La commission n'a pas souhaité remettre en cause la philosophie du droit en vigueur, qui repose sur un régime d'opposition expresse, maintenue d'ailleurs par le texte transmis par l'Assemblée nationale.

Le régime d'garantit aussi, je le rappelle, la pérennité d'un secteur économique qui emploie directement aujourd'hui plus de 56 000 personnes en France. En revanche, la commission a jugé indispensable de renforcer davantage les mécanismes de régulation déjà présents dans notre droit

à compter du 1 août 2019, dans le cadre du nouveau plan de numérotation de l'Arcep, il sera interdit d'appeler depuis l'étranger avec un numéro géographique national,

une mesure de simplification pour les consommateurs, notamment les plus vulnérables. Il faudra toutefois être attentif aux modalités d'identification du consommateur par la voie téléphonique. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement. il tend à intégrer aux clauses obligatoires des contrats de téléphonie listés à l'article L. 224-30 du code de la consommation l'information du consommateur de son droit de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. J'émets également un avis favorable sur cet amendement, qui me semble positif pour renforcer l'information du consommateur sur ses droits.

Le scrutin est ouvert.

apparaît superfétatoire, d'autant qu'une telle exigence pourrait retarder l'entrée en vigueur de ces chartes. Le présent amendement vise ainsi à rétablir le texte adopté par les députés. L'amendement

Toutefois, dans la mesure où la fixation de ces normes déontologiques est renvoyée à l'adoption d'un décret, il est utile de préciser qu'elles doivent comprendre, sans s'y limiter, des dispositions encadrant les jours et les horaires où les appels sont autorisés,

que les professionnels du démarchage téléphonique devraient respecter sous peine de sanction administrative. Or le dispositif proposé par la commission des lois me semble plus opérationnel et rigoureux que celui adopté par l'Assemblée nationale. Il paraît donc mieux répondre à vos attentes, ma chère collègue. Je m'explique. Le texte de la commission prévoit la définition de normes déontologiques par un décret qui serait pris après consultation du Conseil national de la consommation.

: La parole est à Mme Sylvie Vermeillet. Le démarchage à des fins commerciales sur les téléphones cellulaires est de plus en plus fréquent. Or, contrairement aux numéros des téléphones fixes, qui sont publics ou à la portée de tous dans différents annuaires, les numéros des téléphones cellulaires restent privés. Lorsque le démarchage à des fins commerciales s'effectue sur des téléphones cellulaires, c'est à l'insu et sans le consentement de leurs détenteurs. Cet amendement vise donc à interdire le démarchage sur les téléphones cellulaires.

précisément en train de confirmer, de conforter même, pour les consommateurs. En outre, il existe sur les téléphones mobiles des dispositifs plus protecteurs que sur les téléphones fixes, une option permettant notamment de « bloquer » tout appel jugé indésirable.

le démarchage sur les téléphones mobiles représente une très forte proportion de l'activité de prospection commerciale, car, vous le savez bien, de moins en moins de personnes ont une ligne fixe. En témoignent les dernières données de l'observatoire de l'Arcep s'agissant du trafic de téléphonie

voté avant l'heure où je serai obligé de lever la séance. Peut-être que, lorsque les arguments sont les mêmes, notamment les avis du Gouvernement et de la commission, on peut restreindre un peu plus les explications de vote ... C'est un conseil, pas un ordre. L'amendement n° 33, présenté Le Gouvernement souhaite renforcer le dispositif d'opposition au démarchage téléphonique en vigueur et entend s'assurer du strict respect par son gestionnaire, la société Opposetel, des obligations légales et contractuelles qui lui incombent à travers l'action de contrôle de la DGCCRF. Il convient en conséquence de privilégier la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport d'évaluation de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Quel est l'avis de la commission ? Le présent ? Le présent amendement tend à supprimer l'obligation, introduite par la commission des lois, faite à l'organisme gestionnaire de la liste d'opposition au démarchage téléphonique de rendre accessibles, sous un format ouvert et aisément réutilisable, les données essentielles de son activité. Nous avons souhaité créer un régime de publication en, afin notamment de permettre au Gouvernement, au Parlement, au Conseil national de la consommation et aux associations de consommateurs de mieux contrôler l'action de l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Nous avons rejoint nos collègues députés ainsi que les associations de consommateurs sur la nécessité de disposer de davantage d'informations sur l'activité de l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage téléphonique, notamment pour s'assurer de son efficacité et pour mieux définir ses priorités.

vous connaissez la position de la commission des lois sur les demandes de rapport au Gouvernement : telle n'est pas, selon nous, la façon la plus efficace pour le Parlement d'effectuer son travail de contrôle. De manière générale, de telles mesures procèdent le plus souvent d'une simple volonté d'affichage,

d'exercer son simple rôle de délégant et tout moyen, donc, de demander à son délégataire toute information utile permettant de vérifier la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. donc vraiment étonné : il s'agit presque d'une affaire interne à l'État ; c'est à lui d'exercer, tout simplement, son rôle de contrôle sur la mission qu'il a déléguée.

Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui a introduit pour des manquements en concours un plafonnement pour l'exécution cumulative des amendes administratives prévues par le code de la consommation, ainsi qu'en cas de cumul de sanctions administratives et pénales. Le plafonnement pour l'exécution cumulative des amendes administratives prévu par l'article 3 ne se limite pas- c'est un point important -aux seules sanctions applicables en cas de manquement aux règles relatives à l'opposition au démarchage téléphonique. Il s'applique également à la mise en oeuvre de l'ensemble des sanctions administratives prévues par le code de la consommation. Autrement dit, le plafond qui est introduit ici empêchera de sanctionner cumulativement non seulement un problème lié au démarchage téléphonique, mais d'autres infractions au code de la consommation qui pourraient être bien plus graves et bien plus préoccupantes pour le consommateur.

nous avons rétabli la règle de plafonnement des sanctions administratives en cas de manquement en concours, c'est-à-dire lorsqu'ils sont poursuivis en même temps, lors d'une même procédure ou de procédures séparées. Le droit en vigueur depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 prévoit que les amendes s'exécutent cumulativement. Cela pose question au regard du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, compte tenu

est susceptible de se poser de manière récurrente. En matière de démarchage téléphonique, le manquement peut se répéter autant de fois que le professionnel appelle en numéro masqué ou méconnaît l'interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Si l'administration est bien sûr tenue, dans son pouvoir d'appréciation, de respecter le principe de proportionnalité, je rappelle que l'exigence de proportionnalité s'impose tant à l'auteur d'un texte édictant une sanction- en l'occurrence, législateur -qu'à celui qui inflige une sanction pour réprimer un manquement particulier. Le texte de la commission, dans son 1°, prévoit donc que les sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé. En second lieu, le texte de la commission, dans son 2°, rétablit la règle plafonnant le cumul d'une amende administrative et d'une sanction pénale, en cas de sanctions infligées à raison des mêmes faits, qui ne figure plus dans le droit en vigueur.

se poser lorsqu'un professionnel méconnaît l'interdiction de contacter un consommateur inscrit sur la liste Bloctel, ce comportement pouvant aussi être incriminé au titre de l'infraction délictuelle punie, à l'article 226-18-1 du code pénal, de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, réprimant le « fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne,

aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l'objet d'un contrat en cours. Il tend à remplacer la formulation actuelle, qui interdit la sollicitation des personnes inscrites sur la liste Bloctel, « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes

On peut déjà s'étonner que cette exception existe. Un consommateur qui fait la démarche de s'inscrire sur la liste Bloctel n'a sûrement pas conscience que, dans certains cas, il pourra être sollicité par téléphone, Aujourd'hui, le code de la consommation prévoit qu'un consommateur ayant « des relations contractuelles préexistantes » avec le professionnel peut être démarché, même s'il est inscrit sur la l'article 5, les députés, avec le soutien du Gouvernement, ont restreint cette exception aux seules « sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ». Cette rédaction nous semble équilibrée. En rester au droit existant, comme nous le propose notre rapporteur, participera à n'en pas douter au sentiment que Bloctel fonctionne mal, puisque, même en s'y inscrivant, le risque de démarchage reste très important.

s'agissant de « l'exception client », laquelle permet à un professionnel de démarcher un consommateur même s'il est inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ces amendements visent à restreindre le champ des sollicitations possibles aux hypothèses où le consommateur a un contrat en cours d'exécution avec le professionnel, la sollicitation devant avoir un lien direct avec l'objet dudit contrat.

Ce faisant, ces amendements tendent à revenir sur la position de la commission, qui a préféré en rester au droit en vigueur prévu à l'article L. 223-1 du code de la consommation. Cet article permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des « relations contractuelles préexistantes La restriction du champ d'application de l'exception client que tendent à prévoir ces trois amendements pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. C'est important introduirait d'ailleurs, de fait, une distorsion liée à l'activité économique. Dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d'un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu'ils souscrivent avec le consommateur- contrats à exécution successive. Dans d'autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception. À cet égard, la CPME nous a indiqué que cette distorsion concernait particulièrement les commerces de proximité, qui, pour la plupart, n'ont pas de contrat en cours avec leur clientèle, mais souhaitent leur proposer de nouveaux produits.

qui signalent un numéro dans l'annuaire inversé des numéros de services à valeur ajoutée, géré par l'instance d'autorégulation du secteur, le font de leur propre de leur propre initiative, par volonté d'aider l'administration. Les signalements recueillis sont indispensables à l'autorégulation ainsi qu'à l'efficacité des contrôles à visée répressive menés régulièrement par l'administration. Ils permettent d'identifier les auteurs et les techniques de fraude. de déposer un signalement ne donne droit à aucune compensation d'un éventuel préjudice. C'est un acte citoyen du consommateur, et seule une infime minorité de victimes prennent le temps de signaler les numéros frauduleux.

Jomier. L'article 8 prévoit une exception à la publication des sanctions dans le cas d'un préjudice grave et disproportionné. Cet amendement vise à s'assurer que cette exception sera mise en oeuvre uniquement dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique et incluant des données personnelles. Il ne faudrait pas que n'importe quel préjudice grave et disproportionné, tel qu'une baisse de chiffre d'affaires ou une atteinte à la notoriété d'une marque, puisse relever de cette exception. S'il est adopté, cet amendement permettra de garantir l'efficacité du principe de publication des sanctions instauré par l'article 8.

Dans les faits, beaucoup d'entreprises de démarchage vendent en permanence des produits en promotion. Le consommateur est ainsi dupé par un prétendu rabais, qui n'est pas limité dans le temps et qui n'est

Cet amendement tend à interdire les opérations promotionnelles hors soldes lors d'un démarchage téléphonique. En premier lieu, premier lieu, tout type de vente répondant aux critères édictés par l'article L. 310-3 du code de commerce régissant les soldes entre dans le champ d'application de cet article, y compris le démarchage téléphonique. Il ne peut donc absolument pas être fait référence au terme « soldes » en dehors des conditions prévues par la loi. En second lieu, je ne vois pas à quel titre on interdirait la mention d'éventuels rabais hors soldes proposés dans le cadre d'un démarchage téléphonique si ces rabais peuvent être proposés pour d'autres types de vente.

n'hésitaient pas à faire du démarchage auprès des personnes touchées par un deuil afin de vendre leurs produits. Et il n'y a quasiment aucune poursuite judiciaire ! Une nouvelle entreprise propose

par des prestations annexes discrètement proposées en ligne, comme la livraison de fleurs ou l'impression d'un recueil de condoléances. Cette entreprise a passé, en toute impunité, un partenariat avec un grand quotidien du matin, dont la rubrique nécrologique est particulièrement connue. Une famille qui publie un avis de décès dans ce journal se voit donc créer systématiquement, et sans aucun accord de sa part, un espace privé dédié au défunt. De nombreux témoignages ont été recueillis. Par exemple, M. X est décédé à soixante-quinze ans, un mardi. Lors du rendez-vous au service catholique des funérailles, ses deux enfants ont eu la surprise de découvrir, sur l'écran du conseiller funéraire, une page créée au nom de Nicolas, avec sa photo, ses coordonnées, la date et le lieu de ses obsèques. La famille indique alors qu'elle n'est pas intéressée par le service proposé. Pourtant, un mail est adressé aux enfants avec le lien vers cette page et, le lendemain du décès, la fille du défunt reçoit un appel sur son portable pour la relancer et pour savoir si le service a bien été proposé.

ferme, mais totalement inopérante. Je voulais, grâce à cet amendement, attirer l'attention du Gouvernement sur ce problème. Depuis des années, les services de l'État sont totalement défaillants. J'ai cité une entreprise qui a passé un partenariat avec un grand quotidien national

Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 et à celles de l'article 56 de la Constitution, la commission des lois a fait connaître qu'elle a émis, lors de sa réunion de ce jour, un vote favorable, d'une part, à la nomination de M. François Pillet- 25 voix pour, aucune voix contre -et, d'autre part,

Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, présentée